La séance est reprise et l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État et article 41 bé du projet de loi de finances, la parole d'abord à Madame Isabelle briquet, rapporteur spécial de la commission des finances. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la promesse du gouvernement de réarmement de l'État territorial trouve une traduction budgétaire d'une ampleur très limitée, en effet, les effectifs de l'administration territoriale de l'État augmenteront en 2023 de 48 équivalents temps plein, soit une hausse de seulement 0 16 % peut-être s'agit-il de l'amorce d'un changement de paradigme, mais en tout état de cause, c'est une avancée bien limitée au regard des enjeux considérables de la mission, je souhaite aborder dans un 1er temps les grands enjeux de la réforme de l'organisation territoriale de l'État, les préfets sont au coeur de cette réforme, et singulièrement les préfets de région, qui peuvent en fonction des priorités locales et nationales redéployer jusqu'à 2000 équivalents temps plein par an entre missions budgétaires, outre la mission a GTE ces mouvements concerne l'émission agriculture écologique culture travail emploi solidarité économie alors que le bilan des redéploiements avait fait l'objet d'un amendement du gouvernement au projet de loi de finances rectificative, rien n'a été déposée avant la CMP ces situations nuit à l'information du Parlement sur les priorités mises en oeuvre dans les territoires, par ailleurs, les secrétariats généraux communs départementaux rencontrent d'importantes difficultés, cette réforme n'a pas suffisamment été anticipé les chantiers de convergence sur le périmètre de l'administration territoriale de l'État doivent impérativement s'accélérer pour permettre à ses services de fonctionner dans de bonnes conditions, je souhaiterais également aborder les constats dressés par la Cour des comptes dans son rapport sur les effectifs de l'ennemi de l'administration territoriale constat que je partage entièrement la cour considère ainsi que les suppressions de postes de ces dernières années n'ont pas été réaliste au sein des préfectures qui fonctionne, qui ne fonctionnent pardon qu'au moyen de contrats courts qui précarisent leurs titulaires et désorganise les services la Cour fait également le constat que le plan peuvent préfectures nouvelle génération PPNG de 2016 a été conçu pour adapter l'émission réduction d'effectifs et non l'inverse, en 10 ans, le programme a réalisé un schéma d'emplois cumulés de moins 4748 équivalents temps plein, soit plus de 16 pour 100 des emplois au rythme du réarmement annoncé pour 2023, il nous faudrait un siècle pour parvenir à la situation de 2010, le ministère de l'Intérieur a également mis en place un document stratégique mission prioritaire des préfectures 2022 2025, ce document porte mal son nom puisque loin de prioriser l'émission par rapport à d'autres, il se contente de reprendre l'ensemble des missions des préfectures, il est donc nécessaire que l'éclat que l'État clarifie son discours ou bien les préfectures doivent prioriser leurs missions et à ce titre, l'émission les moins importantes auront vocation à abondé en moyens et en emplois les missions prioritaires ou bien aucune mission ne peut, perte d'emploi, ce qui d'ailleurs et mon et mon avis et il faut conforter en urgence les effectifs et les moyens des préfectures par ailleurs depuis plusieurs mois, les délais de tension de carte nationale d'identité et de passeport atteignent les délais inacceptables fin mai dernier, une personne souhaitant obtenir un passeport ne pouvait en moyenne espérer en disposer avant la mi-septembre si le gouvernement à augmenter la dotation de la dotation Titres sécurisés à destination des communes, l'augmentation du nombre de dispositifs de recueil ne me sont pas en phase avec l'évolution des demandes de titres en l'accueil du public et très juin préfecture dont on ne connaît que trop les nombreuses difficultés des renforts en contractuels sont prévus jusqu'en 2024 je regrette le choix de recourir à des vacataires qui laissent penser qu'il ne s'agit que des des renforts ponctuels, alors que la priorité devrait être de consolider les les services et de fidéliser des compétences, le gouvernement fait encore une fois, le choix de recourir à des vacataires, je souhaite évoquer pour conclure, la situation des intervenants sociaux en commissariat de police et en unités de gendarmerie, vous en conviendrez, sans doute, Madame la Ministre, il joue un rôle majeur pour l'accueil des victimes en situation de fragilité femmes victimes de violences intrafamiliales, personnes en situation de handicap et j'appelle de toute urgence à clarifier le régime de financement de ces intervenants alors que l'État se désengage au détriment des associations et surtout des départements, je souhaite que l'État suive au minimum les recommandations d'un rapport de l'Inspection générale de l'administration en stabilisant ses financements à hauteur de 33 % de prise en charge par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance au regard de ces considérations, la commission a émis un avis défavorable sur l'adoption des crédits de la mission. Je vous remercie, la parole est maintenant à Madame Cécile Cukierman, rapporteur pour avis de la commission des lois. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission ah GTE n'appelle pas d'observation particulière en ce qui concerne le programme 232 vie politique la forte diminution de l'ordre de 75 % des crédits s'explique par un calendrier électoral, à ce jour moins chargé en 2023 et le programme de 216 conduite et pilotage des politiques de l'intérieur de l'augmentation, sert à financer la stratégie immobilière du ministère et le renforcement des moyens du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, c'est donc bien la question des moyens alloués au programme 354 administration territoriale de l'État, qui constitue l'enjeu essentiel de cette mission, tant la situation du réseau préfectoral et en 1er lieu celle de l'échelon de proximité, qui représente les sous-préfectures et préoccupante, le projet annuel de performance de la mission Agettes prévoit un véritable réarmement de l'État territorial dans la continuité des missions prioritaires des préfectures 2022 2025 et du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoyait déjà un renforcement des services déconcentrés, je salue la prise de conscience salutaire du gouvernement qui sont désormais comprendre que l'État ne peut pas continuer à diminuer sa présence dans les territoires, au risque d'amplifier le sentiment d'abandon de nos concitoyens comme des élus locaux toutefois ces annonces interviennent après des années de coupes budgétaires drastiques qui ont conduit à la suppression cumulée de 14 % de l'effectif initial de l'administration territoriale de l'État entre 2012 et 2020 et des réformes incessantes qui ont mis à mal les services de l'État, je rappelle que les secrétariats généraux communs départementaux ont été créés au 1er janvier 2021, dans le but de mutualiser les fonctions support des préfectures et des directions départementales interministérielles et de générer des économies, nous n'avons pas encore eu le temps de dresser le bilan de cette réforme que le gouvernement déploie déjà un nouveau plan d'action pour les profs Pictures à horizon 2025, l'annonce de la création de 210 équivalents temps plein sur les 3 prochaines années, l'ouverture de six, sous-préfecture, cette année, dont 5 sont en réalité des des jumelages de sous-préfecture fermée au gré des réformes administratives successives m'apparaissent dérisoires au regard des besoins de l'atrophie qu'a subi l'administration territoriale de l'État depuis plus de 10 ans, ainsi pour l'année 2023, le projet de loi de finances prévoit de revaloriser le schéma d'emplois à hauteur de 48 ETP, soit une hausse certes mais modeste de 0,16 % du nombre d'emplois de même si je salue l'augmentation de l'ordre de 13 % en autorisations d'engagement et 7 % en crédits de paiement, il convient de rappeler que l'impact réel de cette hausse est minorée par la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique, dans un contexte de tensions inflationnistes, dans ces conditions, le réarmement de l'État territorial relève plus de la communication qu'une réelle conviction du gouvernement pour ces raisons, la commission des lois a émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de cette mission. Je vous remercie, dans la suite de discussions, je vous rappelle que temps de parole attribués à chaque groupe pour Jacques unité discussion qu'on prend le texte d'intervention et celui d'explications de vote et le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir, la parole est à monsieur Dominique Théophile pour quatre minutes.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la mission Administration générale et territoriale de l'État, piloté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer verra ses crédits augmenter en 2023 de 18 32 % et de quatre 14 % en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sous l'effet principalement de la hausse du coût de l'énergie d'investissements importants dans l'immobilier et dans le numérique et d'une manière générale du réarmement de l'État dans nos territoires le programme 354 administration territoriale de l'État, qui représente à lui seul 60 % des crédits de la mission pour tous les moyens de réseau préfectoral et des services placés sous l'autorité des préfets de région et les directions départementales interministérielles, il connaîtra en 2023, une hausse de ces crédits de paiement de 13,3 % par rapport à 2022 afin de renforcer de manière inédite, les moyens et les effectifs de l'administration territoriale de l'État, le nouveau schéma d'emplois triennal, plus de 210 TP, dont 48 pour la seule année à venir et, bien sûr, à saluer et à mettre en perspective avec le nombre d'emplois supprimés entre 2012 et 2020, cette évolution traduit, je l'ai dit, le renforcement de la capacité d'action de l'État et met fin à plus de 20 années de réduction systématique des effectifs départementaux et nous le souhaitons à la lente érosion des Liens entre l'État et ses citoyens conformément aux recommandations de la Cour des comptes, un rééquilibrage de la répartition des emplois entre les préfectures devraient par ailleurs être progressivement mises en oeuvre au profit des territoires les plus exposés, je pense notamment à Mayotte, autre motif de satisfaction, le nombre d'apprentis dans le réseau de l'administration territoriale devrait continuer à croître en 2023, rappelons que 622 à apprentis étaient présents dans ce réseau au 31 décembre 2021 il était 2 fois moins nombreux en 2020, enfin, l'Agence Nationale des Titres aussi des titres sécurité l'ANTS verra ses effectifs augmenter pour tenter de répondre aux difficultés rencontrées un peu partout en France dans la délivrance des titres sécurisés, sans surprise, le programme de 132 Vie politique cultuelle et associative qui regroupe les crédits destinés à l'organisation des élections de la Cnccfp et à l'aide publique aux partis enregistrera en 2023 une baisse importante du fait de l'absence d'élections d'envergure au suffrage Direct, notons cependant puisque le sujet nous concerne tout particulièrement que l'organisation des élections sénatoriales de septembre 2023 et des élections territoriales en Polynésie française, nécessiteront que quelque 37 71 millions d'euros en autorisations accord d'engagement en baisse de 79 90 % par rapport à 2022, quelques mots enfin sur le programme de 116 conduite et puis l'autre et pilotage des politiques de l'Intérieur, programme qui porte les moyens et les employes d'une grande partie de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer 96 milliards d'euros en autorisations d'engagement et un vieux 87 milliards d'eau en crédits de paiement, il bénéficiera en 2023 de la plus forte augmentation de crédit en valeur comme en volume, le fonds interministériel de prévention de la délinquance, créée en 2007 sera par ailleurs doté de en 2023 de 84 millions d'euros en autorisation de paiement et un crédit de témoins permettra de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance de sécurisation de la prévention de la radicalisation les commissions des finances et des lois ont estimé, et nous le regrettons que les moyens alloués à cette mission n'était pas à la hauteur des ambitions affichées, je vous propose, à l'inverse de ne pas bouder notre plaisir de réarmer notre État territoriale en adoptant ces crédits et je vous remercie. Merci, la parole est maintenant Madame Florence Béatrice comptable pour 6 minutes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, au travers de la mission à GTA, le ministère de l'Intérieur mette en oeuvre 3 de ses responsabilités fondamentales garantir l'exercice des droits des citoyens : assurer la présence et la continuité de l'État sur le territoire et et mettre en oeuvre au plan local et politiques publiques nationales notre propos portera principalement sur le programme 354 relatif à l'administration territoriale, tout d'abord un constat unanime le retrait de l'État territorial, tout le monde s'accorde à dire que l'État territorial se trouve actuellement dans une phase de recul, comme en témoigne le dernier rapport de la Cour des comptes sur les effectifs de l'administration territoriale de l'État et le récent rapport d'information de nos collègues Agnès Canayer Éric Kerrouche la Cour des comptes constate que l'administration territoriale de l'État a perdu 14 % de ses effectifs en une décennie, et que les baisses subies par les services déconcentrés de déconcentrer sont souvent disproportionnés par rapport à celles supportées par les services centraux, au surplus, alors que les territoires doivent massivement investir dans les transitions, le ministère de l'Écologie a fait le choix de faire peser cette baisse sur les services départementaux au final la Cour juge les suppressions au sein des préfectures irréalistes, elle considère que les schémas d'emplois postérieurs à 2008 mai 2018 mettre à mal le renforcement des missions prioritaires des préfectures d'autant plus que celles-ci ne sont pas définis, le rapport de nos deux collègues Agnès Canayer Éric Kerrouche monte que la chute des effectifs au sein des DDI et de l'ordre de 36 % en 10 ans et de 10 % pour les personnels des préfectures et sous-préfectures, sous-préfectures cette baisse drastique et continue a été compensé par le recrutement de personnels contractuels précaires pour de courtes durées, ceux qui précarisent bien entendu les agents désorganise les services et complexifie la gestion des services, la rapporteure spéciale Isabelle abonde également dans ce sens, mettant en exergue la perte de compétence et donc la perte d'expertise de l'État qui découle de cette stratégie d'économie de moyens, visiblement le gouvernement lui-même partage ce constat, le projet annuel de performance de la mission, indique que l'évolution des moyens dédiés au fonctionnement de l'administration territoriale de l'État, traduit un renforcement de la capacité de l'action de l'État sur le terrain, mettant ainsi fin à plus de 20 ans de réduction systématique des effectifs départementaux, cependant, ces moyens sont en idées équation avec le discours de réarmement des territoires, porté par le gouvernement, quel est au fond la doctrine territoriale de l'État, au vu de ce constat unanime, il aurait été logique que le gouvernement mobilise les moyens nécessaires au renforcement de l'action de l'État dans les territoires, pourtant la hausse présenté dans le projet de loi de finances pour 2023 est en trompe-l oeil, car elle est principalement lié en réalité à l'augmentation du point d'indice et ne permet pas de répondre aux besoins, elle représente en réalité un demi-TP par préfecture et la répartition entre les effectifs y'flou et ne précise aucun critère de détermination des redéploiements, cette situation est d'autant plus préoccupante que la Cour des comptes, a souligné le vieillissement des agents territoriaux, ce qui imposerait logiquement recrutement échelonner au fil du temps développement de l'attractivité dans certaines régions, si le nouveau plan missions prioritaires des préfectures 2022 2025 marque un changement de philosophie, mais on peut le saluer les moyens alloués, peine à convaincre forcé de constater que les délais pour l'obtention des titres d'identité, cela a été dit bon croissant et qu'il en est de même pour les demandes de titre de séjour, les collectivités n'ont toujours pas pu bénéficier de redéploiement d'effectifs en matière de conseil en ingénierie et contrôle de légalité le récent rapport de la Cour des comptes estime que la qualité de contrôle se dégrade, elle est d'autant plus critique que les recommandations formulées en 2016 n'ont pas été suivies d'effet, par conséquent, comme nous l'avons déjà dit les il y a lieu de s'interroger sur la doctrine territoriale de l'État et de faire un choix : soit l'émission des préfectures sont de même niveau et dans ce cas il faut donner à l'administration, les moyens de ses ambitions, soit il faut sélectionner donc clarifier les missions de l'État et renforcer certains postes, or le gouvernement ne choisit pas, et l'État touche-à-tout perdure sans en avoir les moyens, donc il dysfonctionne, nourrissant ainsi un sentiment d'abandon dans nos territoires, alimentant les frustrations qui ont elles-mêmes des effets électoraux délétère, peu de domaines d'action publique ont connu autant de réformes en nombre un cadencement sans qu'une évaluation soit réalisé à chaque étape, il est impératif pour l'état de clarifier son organisation avec ses représentants, comme son rapport aux collectivités territoriales pour rendre l'action publique, lisible et efficace : garantir un service public de proximité qui est le pilier de notre République, s'agissant des 2 autres programmes de la mission budgétaire le calendrier électoral de 2023 réduit à raison les crédits du programme de 132 vie politique les investissements dans le numérique et l'immobilier, traduit par le programme de 116 sont positifs mais d'importants efforts restent à fournir pour les applicatifs utilisés localement de même si la poursuite des investissements en matière de numérique est nécessaire, il reste à évaluer les effets de leur déploiement dans le temps car le numérique représente à la fois un besoin et une limite de l'État territorial pour conclure, si on peut saluer la prise de conscience de l'exécutif sur le nécessaire réarmement de l'État territorial, nous partageons les conclusions de la rapporteure sur l'INA l'inadéquation des moyens mobilisés et voteront donc contre l'adoption de cette mission budgétaire, je vous remercie, merci. La parole est à la présidente : Éliane Assassi pour le groupe CRCE et pour quatre minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je veux dire, je tiens tout d'abord à remercier nos deux rapporteurs dont dont Cécile Cukierman pour leur travail et elles ont, je pense, très vivement rappelé l'importance et la nécessité de la présence de l'État auprès de nos habitants et de nos communes, lorsque j'ai présenté la mission Administration générale et territoriale de l'État en 2021 j'noter déjà une stagnation des moyens alloués à cette mission, aujourd'hui, il est vrai que l'on peut noter une légère hausse mais qui n'est quand même pas à la hauteur des besoins pour compenser les 10 années de désengagement de l'État dans nos territoires, nous devons réaffirmer les territoires, ce qui n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien 1er ministre Jean Castex, la crise des gilets jaunes, suivi de la crise sanitaire ont témoigné des limites de l'État dans nos territoires pendant plus de 10 ans, on a réduit les moyens financiers et humains qui ont eu des conséquences lourdes sur la gestion quotidienne dans les services déconcentrés de l'État, pourquoi un désengagement aussi fort de l'État, où en sommes-nous de cette égalité républicaine tant promis, qui pourtant n'est réel que sur le papier, aujourd'hui ce sont des files d'attente à n'en plus finir devant les préfectures pour renouveler des titres de séjour pour des demandes de naturalisation et j'en passe, il n'y a pas assez d'argent pour accueillir et suivent des dossiers, il n'y a pas un réel accompagnement puisque les méthodes sont imposées d'en haut sans tenir compte des réalités du terrain, les différentes réformes administratives n'ont fait qu'augmenter cette défiance envers les envers les pouvoirs publics, générer des suppressions de postes et fenêtre un mal-être dans votre administration, matelas, des matérialisations, on y revient encore accentue les inégalités et ne permet pas de renforcer la présence de l'État, au contraire, la rationalisation prime sur l'humain et de ce fait un pacte : le service public, nous demandons le redéploiement de l'État sur le territoire et non un semblant de rééquilibrage les maisons France Service qui ont été créés pour accompagner cette dématérialisation témoignent de leurs limites, les Liens sont rompues avec l'administration, les agents n'ont pas la formation adéquate et l'accompagnement de l'usager se heurte à des difficultés d'accès à l'information, c'est une réalité de nos territoires, autant dans les milieux ruraux à l'échelle urbaine et je connais bien le sujet, en Seine-Saint-Denis, ce sont des milliers de gens qui ne peuvent accéder à des services publics pour répondre à leurs problématiques quotidiennes, la défenseure des droits alerte sur cette dématérialisation qui augmente les saisines puisque l'accès au droit, au pluriel est mise en cause encore une fois, ce sont les collectivités territoriales qui supporte ces tas de réforme parfois sans les ressources et l'ingénieur est nécessaire aussi, rappelez-vous, mes chers collègues, les délais d'attente rallongés, il y a quelques mois encore pour obtenir une carte d'identité ou un passeport, ce sont plusieurs centaines de communes qui n'avait pas les matériaux pour la bonne gestion, c'était des délais rallongés en préfecture de traitement de dossiers, faute de personnel pour s'en charger les collectivités territoriales, les élus locaux n'attendent qu'une seule chose : travailler de manière intelligente avec l'État et ses représentants, le préfet du département ou de sous-préfecture doit être en pleines responsabilités dans son territoire, il doit faire avec les élus afin de comprendre chaque réalité territoriale et apporter les réponses nécessaires, le couple mère préfet était si si applaudit si félicité durant la crise sanitaire pour autant le mariage semble encore loin, ce ne sont pas des politiques imposées par l'eau qui permettront d'obtenir des résultats positifs et de ce fait d'améliorer le service public pour les habitants, il faut faire avec celles et ceux en gestion quotidienne parce qu'aujourd'hui il est bien là le problème : on demande aux collectivités d'assumer des missions alors qu'on opère des restrictions budgétaires qui mettent à mal les finances locales l'horizontalité doit être le maître mot pour que l'État renoue avec ses communes et sa population c'est uniquement avec plus de moyens humains et financiers qu'on pourra réarmer les territoires et donc lutter contre l'isolement d'une partie de nos usagers, donc pour toutes ces raisons, je pense que vous l'avez compris, nous ne voterons pas cette mission. Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste et pour six minutes. Mais la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des finances, le président de la commission des lois, mes chers collègues, j'évoquerai 2 points dans cette mission, la fraude documentaire, madame la ministre, fait partie des sujets extrêmement importants et ça concerne cette mission pour ceux qui par pudeur ou par dogmatisme s'évertuent à nous expliquer qu'il n'y a pas de fraude documentaire, je souhaite vous raconter une petite histoire, un individu fiché S, chef d'un réseau sophistiqué de faussaires. Faux papiers d'identité, comptes bancaires usurpées escroqueries auprès automobile a détourné au moyen de 73 fausse identité 193 véhicules alors qu'il était mis en examen depuis 2010 et ce dans le cadre d'une affaire de financement du terrorisme, toujours au sujet de la fraude documentaire je me permets de vous lire ce petit courriel assez récent adressé par le responsable d'un commissariat de l'Orne à l'Association des maires de ce département, par le biais de ce miel, je souhaite vous sensibiliser sur le point suivant, lors de la demande de carte nationale d'identité en mairie, les usagers présente un certificat de naissance ce certificat de naissance peut être vérifié par les agents via le logiciel qu'au Medec qui est facultatif pour les mairies car très onéreux, ne croyez-vous pas, pas, ben la Ministre qu'il serait temps que la saisine de ce logiciel soit gratuite et je vous indique que lorsque l'on demande notamment lors de la loi de finances, monsieur le président de la commission des finances, on essaye d'amender les dispositifs pour avoir de meilleures communications on se tape un article quarante parce que ça crée des dépenses d'amélioration du logiciel, donc si vous voulez améliorer un logiciel au motif qu'il a un peu de difficultés dans la communication ou dans l'échange de données, vous ne pouvez pas le faire par voie d'amendement parce que ça crée une dépense nouvelle, donc il faudrait quand même que c'est ce type d'amélioration puisse être avec vos services. De façon à ce qu'on puisse, notamment en ce qui concerne les mairies notamment en ce qui concerne la sécurisation des titres d'identité pouvoir améliorer des disques. Positif il y a un certain nombre de de sujets comme ça qui sont vraiment extrêmement utile et qui ne peuvent pas passer par le biais d'un amendement par qu'il constitue une dépense nouvelle et c'est un peu dommage, le responsable du commissariat poursuit les voyous profitent de cette faille pour se présenter dans les mairies de ces communes avec de faux certificats de naissance et une demande de carte nationale d'identité si l'agent de la mairie ne s'assure pas de de l'authenticité du certificat de naissance, le demandeur se retrouve avec une vraie carte d'identité mais une identité frauduleuse, donc vous voyez le le le dispositif ça relève complètement de cette mission et à mon avis, c'est tout à fait réparable. Donc moi je crois. Que ce sujet est extrêmement important et par ailleurs je voulais aussi vous signaler qu'il n'existe toujours pas de formulaires Cerfa pour les actes de naissances en France si le contenu de l'acte de naissance et partout le même chaque mairie émet des documents sur son propre près bien en tête ce qui crée évidemment des facilités pour la fraude, je souhaite donc vous demander, notamment, si vous ne pourriez pas ou si le gouvernement ne pourrait pas utiliser le fonds européen pour la sécurité intérieure, le FSI doté d'un nouveau programme de 98 millions d'euros pour la programmation 2021 2027 destinés notamment à des programmes de lutte contre la fraude documentaire et, surtout, c'est le sujet dont je vous parlais il y a une minute l'interopérabilité des systèmes d'information qui est reconduit, dispose de 98 millions d'euros pour faciliter la lutte contre la fraude documentaire et l'interopérabilité des si des systèmes, c'est bien de ça dont on est en train de parler et c'est bien aussi ça qui favorise la fraude documentaire, c'est le fait qu'on communique mal et qu'on échange mal les données. Donc, je vous demande, Madame la ministre, très officiellement, de bien vouloir vouloir considérer ce fonds européen 98 millions c'est pas complètement rien ça évitera au président de rendre un article 40 et et ça nous permettra d'améliorer les dispositifs et puis bah la ministre, on nous dit que le fichier âgé de rêve est en train de va disparaître au profit d'un autre fichier pour les étrangers en France, peut-être que cela relève plutôt de la mission Immigration, mais c'est quand même dans la rubrique des des titres sécurisés et puis pour la minute trente qu'il me reste, je voudrais vous dire comme chaque année, mais doutes sur le le CIP PDR C PDR le le comité pour la prévention de la radicalisation Nat. Toujours aucune évaluation distribue des fonds par ci par là, sans évaluation dans une période qui est particulièrement critique où certes on parle moins de terrorisme et où le sujet de la radicalisation demeure tout aussi important,

excellent d'ailleurs sur les politiques transversales qui a été arraché de haute lutte dans cette maison, mais qui est un document très utile, un comité scientifique, précisément pour la lutte contre la radicalisation qui s'était réuni 3 fois en 2017 3 fois en 2018 et 6 fois en 2019, ce qui fait une croissance exponentielle, mais je n'ai pas trouvé ni en 2020 ni en 2021 2 réunions, peut-être à cause du Covid. Je ne le sais pas quoi qu'il en soit, mais à la mini-je voulais vraiment attirer votre attention sur ces 2 points, la fraude documentaire et les évaluations du CIP PDR ça me sont vraiment très, très important, je vous remercie de votre attention.

Madame la présidente, madame la Ministre Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, de prime abord, les montants annoncés semblent plutôt satisfaisant, nous observons sur cette mission une hausse au global, les crédits de paiement augmentent comme les autorisations d'engagement, cela traduit une volonté de réforme pluri-tant en matière immobilière que numérique que nous ne pouvons que saluer, je pense en particulier au développement du système de communication des forces de sécurité et de secours de dernière génération, le le réseau radio du futur, il est également annoncé une rationalisation des effectifs qui est attendu, mais qui devra répondre aux besoins réels des territoires car voilà le vrai sujet : comment faire pour que nous cessions comme c'est hélas le cas chaque année, l'examen de cette mission de constater le recul de l'État dans nos territoires, notamment les plus ruraux, comment faire pour cesser d'avoir encore, a dénoncé l'effacement progressif des services publics de proximité, au profit de la dématérialisation et du tout numérique, qui exclut de fait une partie de nos concitoyens de l'accès au service, si nous nous battons dans cet hémicycle pour la liberté des collectivités, la décentralisation, nous nous battons aussi pour une déconcentration efficace et valorisant le travail des préfectures et des sous-préfectures, au service des administrés, chacun a conscience, il faut maintenant traduire cela en actes, alors s'il y a du borne dans la présentation budgétaire de cette mission, j'entends aussi les critiques portées par les rapporteurs, elles traduisent les inquiétudes de nos territoires, nous sortons de 10 années de réduction continue des effectifs, comme l'a très justement souligné la Cour des comptes dans son rapport, nous ne pouvant que nous réjouir d'observer que l'année 2022 marque la fin de cette trajectoire avec une stabilisation des emplois, il faudra continuer à s'inscrire dans la durée, nous le souhaitons, du point de vue du personnel, il faut, par exemple, cesser de recourir aussi à des contrats courts est par essence précaire du point de vue des institutions nous, regrettant que ce ce phénomène de multiplication des agences aussi spécialisés qu'éloigné des administrés, lesquels ne parviennent plus à trouver d'interlocuteurs, la délivrance des titres sécurisés et sans doute l'exemple le plus criant de l'échec des stratégies successives visant à rationaliser et mutualiser ce qui n'est pas toujours efficace est synonyme d'économies nous parlons ici de quelque chose qui affecte très concrètement le quotidien des Français et qui par la même occasion continuent de propager les clichés qui entourent notre administration lenteur millefeuille paperasse complexité tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage, hein, qui pourra lui raconter ses déconvenues lorsqu'il a voulu se voir délivrer un document pour l'anecdote, j'ai eu la curiosité de contacter un avocat spécialisé dans les recours en cas de carence de l'ANTS il a eu le loisir de me faire la liste des décisions des juges administratifs enjoignant à l'agence a délivré sous astreinte des permis de conduire, suite à des retards de plusieurs mois en conclusion et suite à ces constats, le groupe RDSE s'abstiendra sur le budget, le budget de cette mission à vous remercie Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est le même marteau qui frappe et on a raccourci le manche affirmer il y a près de 2 siècles, cette image du rôle des préfets comme acteur de proximité de l'État est toujours d'actualité, le préfet et le bras armé de l'État territorial, il incarne l'État au plus proche des administrés, le débat sur l'État territoriale les services déconcentrés, la décentralisation est ancien à mesure du mouvement de décentralisation impulser dans les années 80 l'administration territoriale de la République a évolué avec l'émergence des cons, des collectivités territoriales, cette consécration fait apparaître le lien indéfectible entre l'État et ses services déconcentrés, d'une part et les collectivités territoriales d'autre part, la bonne santé du partenariat, collectivités, État aujourd'hui consacrés par le couple mère préfet conditionne la qualité des politiques publiques, l'exercice des droits et la bonne gestion des ressources publiques au profit des citoyens aujourd'hui nous examinons la mission budgétaire de l'administration générale territoriale de l'État, composé de 3 programmes cette mission budgétaire est en hausse globale mais de manière inégale, cette augmentation n'est pas véritablement à la hauteur d'un réarmement de l'État dans les territoires comme l'appel notamment de ses voeux, notre collègue rapporteur excellente pour avis de la commission des lois, Cécile Cukierman la bonne réception de ce constat effectué depuis plusieurs années sur les bancs de la Haute Assemblée de bonne augure toutefois les moyens nouvellement néfastes toujours pas une décennie de recul de l'État dans les territoires, en effet, les sous-préfectures ont perdu un quart de leur effectif physique entre 2012 et 2019 alors que les besoins ne cessent de s'accroître cet effort salutaire ne sont pas suffisants et au-delà de la simple inscription budgétaire, la réflexion doit aujourd'hui porter sur le rôle même de l'État territorial comment rompre avec le sentiment d'abandon des agents et des usagers et rétablir la confiance en un État territorial performant, comment mieux associer les élus de terrain aux transformations et leur redonner de la lisibilité sur l'action de l'État dans les territoires, comment donner une cohérence à l'enchevêtre ment des réformes successives jamais évalué et toujours empilées les unes après les autres, avec mon collègue Éric Kerrouche nous avons récemment rendu un rapport d'information au nom de la délégation aux collectivités territoriales, dont le titre est signifiant à la recherche de l'État dans les territoires, se fondant sur une large consultation tant d'élus des territoires que des agents de l'État, nous avons étayer ce que nous déplorons depuis longtemps au Sénat une succession de réformes administratives depuis 15 ans qui transforme sans inclure suffisamment les acteurs concernés, plus de 4 élus sur 5 estime ne pas avoir été suffisamment associés aux dernières réformes des services déconcentrés de l'État, de même 43 des préfets et sous-préfets consulté ont le même sentiment, le diagnostic est cinglant : l'État est à la peine face aux attentes des élus locaux, la moitié des mères de moins de deux mille habitants estime que l'offre de service public sur son territoire est défaillante, un nombre croissant de communes se tourne vers les départements vers l'intercommunalité ou le secteur privé en matière d'ingénierie territoriale alors avec Éric Kerrouche nous recommandons plusieurs réformes d'abord d'entrer véritablement le préfet au coeur de l'État territorial la crise sanitaire a souligné les bénéfices du groupe: maire, préfet, il est nécessaire que le préfet connaissent son territoire en y restant plusieurs années et qu'il dispose en période de crise de l'ensemble des services de l'État et surtout qu'il soit le délégué de toutes les agences de l'État, nous pensons aussi qu'il est nécessaire d'instaurer une relation de confiance avec les élus locaux, avec plus de transparence, notamment dans l'attribution des subventions et dans l'évaluation des préfets par les maires, il faut véritablement garantir les moyens de l'État dans les territoires pour qu'il soit plus adapté à une meilleure répartition des effectifs, sortir de la logique systémique des appels à projets et renforcer les moyens, notamment du CM1, enfin il faut assurer une présence territoriale adaptée avec une permanence physique garanti dans les locaux des préfectures et des suppressions sous-préfecture pour lutter contre la fracture numérique, il faut refondre les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité du service public, nos territoires mérite considération moyen et performance, il n'y aura pas de bonne décentralisation sans rhume d'une réelle déconcentration des services de l'État au service des élus et des administrés le budget que nous examinons n'est pas tout n'est pas encore sur cette trajectoire, c'est pour ça que mon groupe le votera pas. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission des lois, les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État que nous examinons ce soir soutiennent ce qui est au coeur de aux institutions républicaines, ils sont en augmentation de 10,32 % l'autorisation d'engagement et 4,14 % en crédit de paiement pour autant, cette hausse des moyens qui intervient après 10 ans de recul de l'État au sein des territoires apparaît insuffisante au regard des enjeux considérables de la mission, le réseau préfectoral est indispensable, notre pays au service rendu à nos concitoyens, or l'administration territoriale de l'État est actuellement très affaiblis par les réformes qui se sont succédés et nous devons faire face à un recul des services publics, surtout des services de proximité, le plan préfectures nouvelle génération mise en oeuvre entre 2016 et 2020, a été fortement orientée sur la dématérialisation des formalités administratives et a profondément remodelé la délivrance des titres tels que les pas ce port les cartes nationales d'identité ou encore les permis de conduire de nombreux points de contact qui permettaient à une population souvent âgés, ou il y pas accès à Internet de disposer d'un interlocuteur dans ses démarches administratives ont été supprimés à autre les publics fragiles se totale absence de mobilité dans un certain nombres de territoires si l'entrée du numérique dans des procédures apparaît nécessaire au vu des évolutions technologiques, la fracture numérique territoriale et sociale ne doit pas être aggravée, or les suppressions successives des relais physique de l'état dans les communes au profit de services en ligne ou trop éloignés, on crée un véritable sentiment d'abandon des habitants des territoires ruraux, même l'implantation des maisons France ce service un peu partout sur le territoire ruraux connaît un succès encore mitigé, il faudra t'évaluer ce concept dans quelques années et surtout poursuivre les financements d'État quant au financement, aujourd'hui des maires se pose les questions, cette réalité, nous la connaissons tous dans les départements ruraux, de même, nous sommes tous confrontés aux retards de de délivrance des titres, les délais d'obtention des cartes nationales d'identité de passeport sont devenues inacceptables pouvant aller jusqu'à 4 ou c'est moi la révolution numérique a ses limites et des moyens j'humain reste est indispensable, je veux enfin attirer votre attention madame la Ministre, sur une autre réalité : la diminution de la qualité de l'ingénieur il territoriale délivrés aux communes, les départements ont souvent pallié la baisse des moyens de l'administration territoriale de l'État en créant des structures chargées de répondre aux besoins des communes en leur apportant soutien et conseils en Aveyron Le département ainsi créé à Véro ingénierie afin d'offrir un accompagnement personnalisé, une assistance administrative, juridique, technique et financières aux collectivités locales et à leurs groupements dans l'exercice de leurs compétences et la réalisation de leur projet, en l'occurrence la charge de cet ingénieur, incombe désormais aux départements et nous on allait et non à l'État, madame la Ministre, chers collègues, la présence de l'État dans les territoires, aux côtés des citoyens, c'est des élus locaux et plus que jamais nécessaire si l'on peut se féliciter d'une prise de conscience du gouvernement sur la nécessité de mieux assurer cette présence territoriale, en revanche, ce budget ne semble pas à la hauteur des enjeux pour cette raison, la majorité du groupe, les indépendants s'abstiendra de le voter.

Madame la présidente, madame la ministre, mesdames les rapporteures mes chers collègues, Madame la Ministre, l'ancien maire d'Arcueil souffrent pour ses sous-préfet au moyen rabougrie et encore plus pour les usagers de ces sous-préfecture, c'est sans doute le cas de nombreux maires et ancien maire, peut être même à Beauvais ce budget présente une augmentation très légère mais peu signifiantes. Depuis 2010, 11763 OPT ont été supprimés dans l'administration territoriale et 4748 dans le réseau des préfectures, soit 14 % des effectifs initiaux et même 24 % pour les seuls sous-préfecture, la commission des lois a souligné que les moyens mobilisés ne sont pas suffisants pour atteindre cet objectif de renforcement de l'administration territoriale de l'État et qu'il est nécessaire de s'interroger en profondeur sur le rôle de l'État dans les territoires, ce que le gouvernement se refuse encore à faire, préférant multiplier des réformes administratives, une traduction concrète et la création des secrétariats généraux communs, ces nouveaux services déconcentrés interministérielle placée sous l'autorité du préfet, mettant de fait des administrations comme celle du ministère de la transition écologique sous sa tutelle, lui-même étant sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, cette organisation nous interroge particulièrement d'autant plus que nous ne sommes pas certain que les premiers retours face éteint fasse état de gains issus de cette mutualisation notre expérience des territoires montre des failles dans l'ambition du fameux couple mère préfet la commission des lois, rappelé d'ailleurs ce problème majeur, les élus locaux ne peuvent compter que sur la bonne volonté des sous-préfets qui entretiennent de plus en plus difficilement une connaissance fine du terrain et un lien de proximité avec les maires de leur arrondissement aussi, nous avons accueilli avec intérêt le début des réouverture des sous-préfectures et le début de renforcement réel d'effectifs, le plan préfectures nouvelle génération 2022 du mail 2025 2025 marquera-t-il un progrès réel, nous le souhaitons, défenseur d'une égalité dans l'accès au service public, je rappellerai que notre groupe n'a cessé d'alerter sur les dangers d'une dématérialisation massive comme seul indicateur d'une modernisation au service du citoyen, l'illectronisme est une réalité qui touche 13 millions de nos concitoyens et chacun d'eux d'entre nous a eu plusieurs expériences vécues ou rapporter de difficultés et de situations délicates, voire ubuesques liées à la fin de l'accueil aux guichets, nous saluons donc le début de l'augmentation attendue d'effectifs d'agents titulaires consacré aux missions d'accueil dans les 3 prochaines années, nous espérons que ce redémarrage pourra aussi servir dans la gestion des titres de séjour à la veille d'un débat ici sur la réforme annoncée de l'asile et d'immigration, nous serons vigilants à ce que la dégradation dans les délais de rendez-vous en préfecture ou de traitement par exemple ne serve pas de justificatif à une aggravation de la situation des étrangers dans leurs Liens et échanges avec l'administration, il est à noter que la commission des finances, a très justement pointé du doigt que la défaillance de l'État dans la délivrance des titres était inacceptable, nous comprenons la diminution des crédits sur le programme, vie politique au regard du ralentissement du calendrier électoral en 2023 nous regrettons l'absence de la démocratie locale et participative dans ces crédits en résumé des aller-retour contradictoires sur la politique d'accueil de l'usager des moyens inadaptés à des réformes dans l'évaluation demeure à faire le recours trop important contractuels dont la pérennisation des emplois et pourtant indispensable notamment pour les intervenants sociaux au coeur du dispositif de prévention de la délinquance Merci, la parole est maintenant à monsieur François Bonhomme dernière orateur pour le groupe Les Républicains et pour cinq minutes. Madame le Ministre messieurs, madame, le rapporteur, mes chers collègues, nous voici donc parvenus à l'examen des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État naturellement cette mission se concentre sur la situation du réseau préfectoral et en 1er lieu assez de l'échelon de proximité que représentent ces sous-préfecture. Maintes fois il a été affirmé votre intention de réarmer l'État territoriale en vous inscrivant dans la continuité des missions prioritaires des préfectures 2022 2025 cette volonté affichée doit s'inscrire hein sa triple mission des préfectures qui ont été rappelés précédemment par les orateurs, car beaucoup avant nous ont regretté que la perte de la présence et de l'efficacité de l'État sous sa forme territoriale qui a beaucoup perdu du terrain ces dernières années au fur et à mesure des différents plans d'action à réforme : la création des secrétariats généraux, communes, départements, de tout, il a près 2 ans est trop récente pour en mesurer les pleins effets en tout cas les effets escomptés : évaluer la réalité et l'objectif de mutualisation des fonctions de support des préfectures et des directions départementales interministérielles ainsi que de créer des économies, je sais que l'annonce, c'est la succession de pannes d'action n'arrange pas les choses, je me demande même si ce n'est pas devenu une sorte de stratégie de communication, néanmoins il y a une chose sur lequel nous y voyons clair c'est les effectifs de l'administration du territoire de l'État, nous pouvons dire que nous sommes à la croisée des chemins : la réforme territoriale de l'État de administration territoriale engagée de la plus de 10 ans s'est traduite par une réduction ininterrompue d'effectifs, c'est quand même une perte de plus de 11000 équivalents temps plein, que nous avons enregistré, soit 14 % de l'effectif initial, ce n'est que cette année que cette baisse a été stabilisé et cette trajectoire interrompue, naturellement, il n'est pas si surprenant que domine un sentiment d'abandon et de perte de présence humaine dans les réseaux des préfectures et même dans l'hypothèse, vous prendriez un soin particulier dans l'allocation des moyens humains et des effectifs en tenant compte de manière fine du niveau d'activité des préfectures ou essayer, préfecture, cela se traduit inévitablement par un effet à neuf assommant accrue de la présence de l'État, que les suppressions de postes dans les préfectures ont manqué de discernement, faute d'analyse adapté, nous avons tous des retours de d'expérience des services au sein des préfectures qui ne fonctionne pas ou mal et, désormais, au moyen de contrats courts de contractuels source souvent nos fragilités de provisoire et de désorganisation des services, il a manqué sans doute une véritable réflexion globale préalables et une analyse plus fine à chaque niveau de service sur la répartition de l'effort en fonction de la réalité des besoins de chaque région, nous avons été un certain nombre à constater, a regretté que dans les directions départementales interministérielles dans certains ministères, je pense celui évidemment de l'écologie et des ministères sociaux a regretté aussi que les suppressions portent sur leurs services départementaux au bénéfice le plus souvent des directions régionales qui ont été largement elle épargnée. Plus structurellement il a la question lancinante et parfois criantes pour l'État qui se heurte au manque d'attractivité de certaines fonctions de certains territoires, je ne vois pas aujourd'hui de stratégie d'ensemble nouvelle ni les moyens suffisants dans cette mission pour en faire en sorte que les postes soient préservés et qui ne reste pas vacants faute de candidats dernièrement la Cour des comptes à formuler des recommandations ceux si je n'y reviendrai pas, mais je pense qu'elle pourrait naturellement nous inspirer, elle vous rend en tout cas, également un guide méthodologique pertinent qu'il revient désormais au ministère de l'Intérieur, de s'approprier et de mettre à l'oeuvre, hein, sa qualité de chef de file d'administration du territoire de l'État. Nous attendons donc un rééquilibrage des emplois entre préfecture en fonction des réalités et des besoins de chaque région, il semble que vous envisagez la création d'un observatoire des effectifs de l'ATE afin de fiabiliser les données relatives aux emplois tant au niveau régional que départemental, qu'en est-il vraiment, on aimerait bien vous entende là-dessus, une chose est sûre, c'est que toute décision doit se faire à Londres d'un principe, c'est celui du rétablissement du lien de proximité, notamment en redonnant au service, les moyens de fonctionner en les rendant plus accessible et en veillant à maintenir un haut degré de qualité autant de principes qui j'espère trouveront une consécration à l'échelle de nos territoires, je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre les excuses de Gérald Darmanin, qui regrette de ne pouvoir vous présenter lui-même ce texte car il est actuellement en déplacement à Bruxelles pour le Conseil Justice et affaires intérieures, la mission Administration générale et territoriale du projet de loi de finances, qui vous est soumis aujourd'hui permet la mise en oeuvre par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de plusieurs de ses fonctions essentielles d'abord, garantir le libre exercice de leur liberté publique par les citoyens, avec l'organisation des scrutins électoraux, assurer une présence continue de l'État sur l'ensemble du pays dans l'Hexagone comme dans les territoires ultramarins et assurer la déclinaison locale des politiques publiques nationales, elle intègre des constantes de l'action ministérielle, mais elle porte également la marque comme la mission sécurité des chantiers d'envergure, portés par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, sur la période 2023 2027, en particulier en terme de réarmement de l'État dans les territoires et de réorientation stratégique du pilotage des politiques de l'intérieur, à l'aune des nouveaux enjeux à relever pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans le contexte de la hausse globale du budget du ministère de l'Intérieur, 25 milliards d'euros pour 2023 la mission Administration générale et territoriale de l'État voici moyen en nette hausse, avec une augmentation de 10 32 pour 100 des autorisations d'engagement et de 4 à 14 % des crédits de paiement, ces chiffres témoignent d'une volonté ambitieuse tournée vers l'avenir et qui se donne les ressources nécessaires pour poursuit ses objectifs dès l'année qui vient plus de la moitié des crédits de la mission sont couverts par le programme administration territoriale de l'État qui témoigne d'un engagement sans précédent pour renforcer la capacité de l'État dans les territoires, partant du constat d'un besoin accru de service public et de proximité de l'État, le président de la République a lancé cette dynamique dès l'an dernier en témoigne notamment déjà l'annonce qu'il a fait le 10 octobre dernier de la réouverture de 6 sous-préfecture : 5 en métropole et une en Guyane, cette évolution qui renverse le courant des 20 dernières années, nécessite de s'appuyer sur des effectifs nouveaux j'oserai vous paraphraser en disant vous voyez nous re-Armon les territoires l'objectif sur 3 ans et de créer 210 équivalents temps plein, 50 pour la seule année 2023, ces créations de postes viennent renforcer les effectifs préfectoraux sur des missions clés, en particulier les services dédiés aux étrangers la délivrance de titres sécurisés qui connaît, comme vous le savez, à fort engorgement en grande partie conjoncturelle, après les 2 années de crise sanitaire ou encore la lutte contre la radicalisation et le terrorisme cet élan de consolidation du réseau préfectoral bénéficiera à tous nos concitoyens en matière de sécurité et de service public, mais aussi aux élus locaux pour la conception et la mise en oeuvre de leur projet et en définitive à l'ensemble de notre pays, nous n'abandonnons pas pour autant les efforts continus menés en faveur de la rationalisation des services de l'État dans les territoires, en particulier en matière de mutualisation étape charnière dans la poursuite de la réforme de l'organisation territoriale de l'État, l'année 2021 a vu la mise en oeuvre des secrétariats généraux communs départementaux, nouveaux services déconcentrés interministérielle placée sous l'autorité du préfet qui permettent de grouper et de rendre plus efficace la gestion des moyens budgétaires des ressources humaines des achats publics ou encore des systèmes d'information et de communication, gage de performances et d'économies leur déploiement se poursuivra pour ce qui est de la conduite, et du pilotage des politiques de l'intérieur, l'objectif constant et celui de la maîtrise des coûts, à la fois en administration centrale et dans les territoires tout en servant la modernisation et l'amélioration des fonctions support indispensable indispensable et je pense en particulier aux enjeux numériques qui constitue une priorité pour l'action du ministère, la direction du numérique se voit attribuer des moyens nécessaires à la réalisation de ses projets d'ampleur comme la constitution du Claude 2ème génération ou encore celle du réseau radio du futur son budget global de 498 millions d'euros sur cette mission doit être mis en regard des autres engagements de la mission sécurité qui prévoit au minimum 381 millions d'euros de dépenses numériques en 2023, notamment pour assurer la transformation numérique des services et l'amélioration des systèmes de communication par ailleurs le ministère poursuit ses efforts de rationalisation de ces emprises immobilières dans l'ensemble du pays afin d'optimiser les coûts et de faciliter concrètement la synergie entre ces différents services de projets sont emblématiques de cette démarche d'abord la création d'un centre unique du renseignement intérieur aujourd'hui répartis sur plusieurs sites qui engage en 2023 43 millions d'euros sur un coût total de 1,3 milliards d'euros, et puis la création d'un grand pôle transversale des directions, support du ministère au-delà, ce sont près de 340 millions d'euros en autorisations d'engagement que le Ministère mobilise afin de permettre notamment la programmation de nouveaux projets d'implantation d'hôtel, de police et de commissariats et 384 millions pour la maintenance lourde du bâti 6 millions d'euros sont aussi spécifiquement dédié pour la rénovation énergétique des bâtiments préfectoraux conformément aux priorités fixées par la première ministre, enfin, ce sont plus de 84 millions d'euros qui sont dédiés au financement de la prévention de la délinquance et de la radicalisation un budget en hausse de plus de 21 % par rapport à l'année précédente, en 2023, ce sera 22 millions d'euros en 2024 24 millions d'euros, le programme de 132 vie politique est le seul qui est en baisse dans la mission, une baisse qui s'explique par le camp de calendrier électoral beaucoup moins chargée, cette année, avec tout de même la tenue des élections territoriales en Polynésie française, ainsi que les élections sénatoriales, mesdames et messieurs les sénateurs, cette mission Administration générale et territoriale de l'État, vous le voyez, va permettre de poursuivre les chantiers de long terme du ministère et de renforcer la présence et l'efficacité de l'État dans tous les territoires, les investissements indispensables à conduire pour faire face aux défis nouveaux qui menace nos concitoyens, il bénéficie de moyens solides, mais il ne s'agit en rien d'une dynamique de hausse de l'ensemble des dépenses en parallèle d'engagement ciblé et conséquent, gage de leur efficacité, la politique de rationalisation et de contrôle des dépenses de fonctionnement se poursuit avec autant de rigueur, j'ai bien entendu, mesdames et messieurs les sénateurs, vos critiques mais ce vous Audrey attirer votre attention sur cet effort historique qui est fait dans le budget de cette mission, jamais le ministère de l'Intérieur n'avait obtenu un tel budget il est néanmoins impossible de rattraper le retard de près de 20 ans de baisse et donc j'espère que ce texte de la chambre en particulier de la chambre des territoires pourra apporter une réponse concrète aux besoins des Français et des Françaises, ainsi qu'aux impératifs de sécurité intérieure, ce consensus, mesdames et messieurs les sénateurs, il vous un parti a désormais de le dégager. Merci. Nous allons maintenant procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État et figurant à l'article premier amendement le 241 monsieur. Merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, cet amendement de mon collègue Guy Bénard vise à augmenter de 15 millions d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement des dépenses de personnel porté par l'action 02 réglementations générales garantie d'identité de la nationalité délivrance des titres du programme 354, les centres d'expertise et de ressources des titres ne disposent pas des ressources humaines nécessaires pour assumer leur mission de manière pérenne, ces défaillances des défaillances ont été analysées par la Cour des comptes dans son rapport public de 2020, après la crise du Covid 2019 les certes on fait face à une multiplication des demandes et n'arrive pas à combler ce retard, une hausse même ponctuel de crédit permettrait sans doute de rattraper en partie ce retard. Merci, est la ville la commission. Merci, le gouvernement a fait le choix d'augmenter sensiblement le le nombre de contractuels au au sein de ces structures ainsi les les demandes de cartes nationales d'identité de passeport alors que ses services compter 35 contractuels en 2021, ils en compte 100 61 ans, je partage avec les auteurs de l'amendement, l'idée qu'il faut pérenniser les emplois au sein des certes et sortir d'une logique de gestion de décrit Sussex successives, hein, alors que l'Agence nationale 10 sécurisé m'a indiqué que la hausse des demandes de titres était durable, il me semble que nous devons avoir pour priorité de recourir à des fonctionnaires titulaires et leur permet de monter de monter en compétence sur leur mission, la Cour des comptes, hein, considère en effet que les préfectures ne fonctionne qu'au moyen de contrats courts et il est important effectivement de titulariser ces postes mais en l'état actuel des choses, je ne pense pas que l'augmentation des crédits proposés au présent amendement permettent de résoudre cette difficulté, il faut impérativement apporter des solutions pérennes au service en question n'ont pas voté des hein des renforts ponctuels pour cette raison, ce sera une demande de retrait. Merci madame la présidente, l'accueil reste en effet une priorité ministérielle, que ce soit dans les préfectures ou dans les sous-préfectures et une partie des 350 créations d'emplois prévues sur la période 2023 2027 et dédiée au renforcement renforcement des c'est compte oh délivrance des titres sécurisés, l'État a renforcé son aide aux communes, avec un budget de de 21 millions d'euros pour pouvoir augmenter le nombre de rendez-vous proposer, aux usagers, qui est une condition évidemment impérative pour diminuer les délais de différence des titres, donc je vous propose soit de retirer cet amendement, sinon ce sera un rejet. Merci, Monsieur Bruillet, vous maintenez

Le plan préfectures nouvelle génération 2022 2025, avait pour objectif le recours massif à la dématérialisation, la fin de l'accueil physique des usagers en préfecture et la mutualisation de fonctions supports, cette politique a eu des conséquences désastreuses, notamment pour l'accueil des publics les plus éloignés du numérique, et pour l'accès au rendez-vous des étrangers dans les préfectures pour ces derniers, il n'est plus possible de se présenter au guichet pour obtenir des rendez-vous pour l'instruction et la délivrance des titres de séjour il il faut prendre rendez-vous par internet et ses prises de rendez-vous sont quasiment impossibles, chaque jour, des personnes se retrouve en incapacité de régulariser leur situation par manquement des services publics, les juridictions font ainsi face à une augmentation très importante des référé mesures utiles pour obtenir des rendez-vous en préfecture en l'absence de créneau disponible sur Internet, la Cimade a ainsi constaté que les ruptures de droit au séjour peuvent être dramatiques pour les personnes concernées, je l'ai constaté moi-même entraînant non seulement un risque d'interpellations en cas de contrôle policier mais causant fréquemment des difficultés dans l'emploi, l'accès à la formation aux études, ainsi qu'aux droits sociaux, le Conseil d'État, dans une décision du 27 novembre

donc à renforcer les moyens humains permettant d'acc médiocre et l'accueil physique en préfecture en par un transfert de 7 millions d'euros. Ce sera là aussi une demande de retrait parce que cet amendement appel de tout de même plusieurs remarques : d'abord le le ministère de l'Intérieur a en partie pris un pris la mesure de l'importance des difficultés les liées à l'accueil des publics étrangers à c'est le choix de renforcer les effectifs quand même à hauteur de 190 équivalents temps plein travaillés par an jusqu'en 2024 en parallèle de la montée en puissance, hein, de que cette évolution doit être accueillie favorablement, même si, comme pour les certains tout à l'heure, la difficulté réside à mon sens davantage dans la pérennisation des postes et la montée en compétence des agents

Je vais donner un petit mot d'explication, madame la présidente, si vous le permettez, je voudrais rappeler qu'entre 2010 et 2020, mesdames et messieurs les sénateurs, les préfectures ont supporté la suppression de 4700 emplois situation que le gouvernement entend corriger désormais désormais depuis 2021 puisque il y a à stabiliser les emplois avec un schéma d'emplois neutre qui a mis fin à ses années de baisse, l'accueil reste donc une priorité ministérielle et une partie des 350 créations d'emplois prévues pour la période 2023 2027 et dédiée au renforcement de cet accueil, ce sera donc même avis que le rapporteur. Oui, un amendement de mon collègue Jean-Pierre de colle le droit de vote et son aboutissement par l'acquisition du suffrage universel est une suite de combats et de lutte acharnée, alors que nous sommes nombreux à prendre conscience de cette conquête acquise au prix de longs sacrifice et de chiffres des élections départementales et régionales de juin 2021 sont tombés comme un couperet : le taux d'abstention était de 65 le 31 % au second tour et de 82 % pour les jeunes, selon les estimations de l'institut de sondages IFOP afin de pallier ce problème démocratique, la proposition de loi numéro 391 déposer un demi de 21 22, déposé par Jean-Pierre de coller ou ateliers proposent de tonton d'automatiser la mise à jour du répertoire électoral unique, le dispositif de ce texte propose que chaque administration communique systématiquement tous les changements d'adresse des administrés à l'Insee pour la mise à jour du répertoire électoral unique sauf mention contraire expresse de l'administrer en conséquence, cet amendement prévoit de créer financièrement un tel programme automatisation du répertoire électoral unique au sein de la mission Administration générale et territoriale de l'État. si je partage le constat des auteurs de l'amendement sur l'exercice du droit de vote et et le souci démocratique qu'il pose, il me semble que la l'amendement proposé impose néanmoins quelques difficultés, il me semble, a priori, qui aurait sans doute un petit souci par rapport au RGPD mais bon, ça c'est à vérifier, et d'autre part, l'automatisation de la mise à jour des informations pour être suffisamment fiables, me semble également complexe à mettre en place, mais peut être là la ministre pourra-t-elle répondre à ce sujet, je pense en enfin qu'il existe probablement d'autres moyens de faciliter les inscriptions des électeurs que de procéder à, à ces évolutions, automatique, je ne partage pas le le principe, ce sera donc une demande de retrait pour ma part. Merci madame la présidente, la mesure proposée par cet amendement de rendre automatique les inscriptions sur les listes électorales des électeurs qui change de résidence, je crois, n'apporterait qu'une solution partielle aux situations de non-inscription et de mauvaise inscription enfin le le citoyen est libre de s'inscrire dans la commune où il souhaite voter et donc cet amendement semble remettre en cause les principes législatifs et réglementaires encadrant la procédure d'inscription sur les listes électorales, d'autre part, je voudrais vous signaler que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer expertise la faisabilité de la mise en place d'un dispositif pour fluidifier la procédure de réinscription, c'est donc un avis défavorable. Je mais vous il retiré merci madame meubles lettre ce contente vous pour le 339. Si madame la présidente, madame la Ministre, cet amendement de ma collègue Martine Filleul, vise à développer les travaux d'intérêt général au niveau local et à lever un certain nombre de freins, l'idée que l'État propose un accompagnement des collectivités territoriales, par une dotation fléchée rattaché au fonds interministériel de prévention de prévention de la délinquance en préfecture le travail d'intérêt général est une peine très intéressante pour certains auteurs d'infractions en ce qu'elle permet de sanctionner, mais également de réparer, voire de réinsérer, elle est une réelle alternative à l'incarcération de courte durée, malgré plusieurs avancées législatives il existe encore dans la pratique des freins à la création de postes de TIG le déploiement de référents TG au niveau local, dont le rôle serait de faire l'interface entre les services d'insertion et de probation et les collectivités et organismes ainsi que le développement de référent visant à faire le lien entre les services pénitentiaires d'un d'insertion et de probation et les services et les services municipaux permettrait la création de postes supplémentaires ce soutien de l'État en direction des collectivités territoriales pour une meilleure réinsertion nous paraît indispensable, c'est pourquoi nous demandons au Sénat de l'adopter, je vous remercie. il me semble, à, à ce sujet qu'il ne faut pas changer la la logique du FIBD qui est d'abord tourné vers la prévention de la délinquance et non pas vers la la sanction ou la la réparation, donc il me semble important de ne pas confondre les dispositifs et de ne pas utiliser le même outil pour prévenir la délinquance et pour la pour la sanctionner, donc les crédits dédiés aux travaux d'intérêt général, sont en effet portées par la mission Justice ce sera donc une demande de retrait. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, moi, je voudrais rappeler que les crédits alloués au FIPD en 2023 sont renforcées, plus 4,81 millions d'euros au regard du PLF 2022 soit une dotation pour cette année de 84,0 9 millions d'euros, ils vont pour permettre de poursuivre le financement de la stratégie nationale de prévention de la délinquance dont, comme vous l'avez rappelé le déploiement des tiges à l'échelle locale alors se présente amendement me semble sans objet, c'est donc à Roger.

au cours des dernières années, la nécessité d'augmenter considérablement la capacité de production de production électrique en énergie renouvelable a pour conséquence un engorgement des services déconcentrés dans les préfectures, l'examen préalable de chaque nouvelle demande d'installation doit suivre une procédure d'autorisation précise mais longue faisant intervenir plusieurs directions et agences, en plus des Dreal qui son chef de file et qui disposent de moyens décentralisée limité à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelables, le Sénat a inséré un article 1er bis visant à créer un référent départemental pour faciliter et accélérer l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition écologique, cette mesure présente l'intérêt de définir un interlocuteur unique en préfecture et par là même de garantir davantage de lisibilité aux porteurs de projet cependant son application risque de se heurter ou sous-dimensionnement des services administratifs par rapport aux flux des demandes, en effet, il ressort des travaux de la rapporteur spéciale au Sénat ainsi que de la rapporteure pour avis de la commission des lois, le constat établi de longue date d'un manque grave de moyens humains au service des services instructeurs dans les départements, sur l'ensemble des territoires et sans moyens en personnel, nous ne parviendrons pas à garantir le déploiement accéléré des énergies renouvelables dans le respect de l'environnement et en cohérence avec les spécificités des territoires d'implantation et vous l'avez bien compris le présent amendement est un amendement d'appel qui me permet de vous interroger, Madame la Ministre, la réalité de l'engagement pris par la ministre de la transition énergétique d'intégrer dans le projet de loi de finances pour 2023, un renforcement des services de l'État. Quel est l'avis de la commission. S'agissant d'un amendement d'appel je vends en demander le retrait mais il me semble en effet indispensable de mieux coordonner les les services de l'État afin de pour mettre la que la multiplicité des intervenants ne fassent pas obstacle aux différents projets Madame la Ministre, je pense que sur ce point là, il faut vraiment faire avancer les choses puisqu'on ne peut pas accepter que sur un sujet aussi important on on est déblocage qui qui freine ainsi considérablement ces projets là. La ministre. Madame la présidente, parmi les missions prioritaires des préfectures pour les années 2022 2025 figure bien l'amélioration de la coordination des expertises, des modalités de suivi des projets territoriaux et

prévues sur la période 23 27 garantissent le maintien des moyens humains dans l'ensemble des services locaux notamment ceux chargés de la coordination des politiques publiques, ça sera donc retrait.

pays de l'Union européenne avoir raté sa cible en matière d'ENR, ce qui lui vaut une amende de 500 millions d'euros, donc nous, nous ne pouvons plus nous permettre d'échouer en matière de développement des ENR et vraiment j'ai des témoignages de, de, de, mettent longtemps à être instruits et il nous faut avancer collectivement sur le sujet, donc je retire mais je serais vraiment attentive au au développement et au suivi de ce sujet. Merci retiré, nous allons procéder au vote des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État,

ils ne sont pas adoptés j'appelle en discussion avec 41 B qui rattache par son examen au crédit de la mission Administration générale et territoriale d'un premier amendement Madame Briquet, au nom de la commission. Très rapidement, madame la présidente, la demande de rapport proposé au présent article porte sur des des évolutions majeures dans les compétences et les moyens de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi la cette commission sur son site Internet, analyse-t-elle le présent article comme un peu à vers une évolution des moyens d'enquête du régulateur financier de la vie politique, même si des précautions ont été prises en en rattachant cette demande aux conséquences budgétaires pour la Commission nationale de telles évolutions, l'objet de la demande de rapport ne relève pas du domaine des lois de finances. Madame la Ministre que l'avis du gouvernement : avis défavorable, je mets aux voix cet amendement de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Je mets aux voix l'article, l'article et donc supprimer, il n'y a plus d'articles et on va donc maintenant passer à l'examen des crédits de la mission Engagements financiers d'État participation financière Accords monétaires compte spécial de près, avance remboursements et dégrèvements.

2 peuchère, c'est à vous. Rapporteur spécial de la commission des finances.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances pourrais presque qui avait appelé chacun, mes chers collègues, il y a tout d'abord une petite remarque pour dire qu'effectivement les conditions, ce débat ne sont pas tout à fait satisfaisant, c'est pas satisfaisant car il s'agit de rien de plus que de parler tout de même de dégrèvement, la plus grosse mission du budget de l'État et juste des charges de la dette, dont on peut estimer que c'est c'est un sujet un peu important, donc c'est quand même un peu dommage de faire ça dans ces conditions, ceci, je tenais à le dire pour que ce soit noté ensuite c'est comme dirait une réclame de notre jeunesse, j'ai quasiment 5 minutes pour vous dire que la mission Engagements financiers de

cette charge d'intérêt qui va grever nos marges de manoeuvre, monsieur le Ministre, notre déficit primaire ne se résorbe pas hé bien, au contraire, nous allons payer des intérêts et des intérêts, alors si en 2022 c'était la mauvaise surprise liée à

hé bien ce ce on, non seulement l'inflation mais également l'augmentation des taux d'intérêts qui ne sont pas terminés, j'écoutais encore, évidemment, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui disait qu'effectivement ce n'était pas terminée, ce Qu'est-ce à dire, ça veut dire qu'en 2023 et encore votre prévision d'inflation est optimiste, hé bien nous allons payer encore plus, et c'est l'effet boule de neige, car notre déficit ne se réduit pas, bien au contraire, en 2023 selon vos prévisions, il augmente encore par rapport à 2022 qui n'aura pas été une si mauvaise année et je le dis sans problème 2022 sera peut-être même encore meilleur que ce que vous avez annoncé et ce que nous avons voté ce matin dans la loi de finances rectificative, nous souhaitons tous, évidemment, pour notre pays, non, il y a encore de de l'effet volume dans cette date et c'est bien ça le problème Monsieur le Ministre, il y avait pas à inverser la courbe de la dette, vous, nous, on ne vous remarquerez d'ailleurs que celui qui avait proposé à un moment d'inverser une courbe s'est pris les pieds dans le tapis, vous faites bien de ne pas le le proposer réellement hélas c'est nécessaire, c'est nécessaire et le FMI que connaît bien aussi Christine Lagarde mais qui, qui n'est plus vous a rappelé à l'ordre lundi où il nous a invités à redresser nos finances publiques rapidement parce que ça ne va plus. Et nous sommes à la veille et l'avant-veille, je crois que c'est le deux décembre alors est-ce que ce sera Austerlitz ou Waterloo on ne sait pas, mais les agences de notation doivent noter la dette française et on verra bien ce qu'ils raconteront sur des perspectives que nous allons avoir, et derrière ces perspectives, ben, c'est évidemment le prix que nous allons payer pour la dette, alors nous avons quand même une chance, il faut le dire, et c'est la force de nos institutions et c'est pas si facile à dire lorsqu'on va parler de charges d'intérêts de la dette, si nous n'avions pas le 49 3. Dans l'état actuel de la démocratie française, sans doute que notre dette serait attaqué par les marchés financiers le 49 3. Bien penser déjà à l'époque, c'est aussi être sûr de pouvoir exécuter un budget. Et c'est important pour un pays comme la France, qui n'a pas fait défaut, c'est ça aujourd'hui la sécurité, alors c'est un petit peu mince et ça ne fait pas une politique totalement construite pour redresser les finances de ce pays dans une large majorité, évidemment pour qu'elle soit bien comprise des Français. Alors nous, nous allons essayer de réduire un tout petit peu le déficit, je ne sais pas si nous vous en tout cas on va vous essayer de vous faire des propositions, et c'est ce que nous avons fait ici au Sénat dans la loi de programmation des finances publiques en à en donnant une nouvelle trajectoire pour essayer de dire allez, si tout le monde fait des vrais efforts on peut arriver aux 3 % en 2025. Mais je crains que ce ne soit pas ce que vous preniez alors Monsieur le ministre, on en parlera tout à l'heure je vais vous faire quelques amendements de propositions car je trouve qu'il a peut-être une incohérence entre les crédits évaluatifs de cette mission et votre scénario macroéconomique, nous en discuterons tout à l'heure. Merci, la parole est maintenant au président rénale qui va d'abord remplacé Monsieur Victorin Lurel, rapporteur spécial de la commission des finances puis le restaurant à la tribune pour remplacer Monsieur Pascal Savoldelli, rapporteur spécial de la commission des finances. La présidente, monsieur le président, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons donc ce soir, les crédits du compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État intervenant comme cela a été dit au nom du rapporteur spécial Victorin Lurel qui n'a pu être parmi nous ce soir, je souhaite réintroduire mon propos par un retour sur la situation du compte depuis 2020, le fonctionnement du compte et très nettement affecté par les conséquences économiques de la crise sanitaire et désormais du contexte international, tant du côté dépenses avec d'importants moyens mobilisés pour aider certaines entreprises du portefeuille que du côté des recettes du fait de l'interruption des cessions d'actifs, il a ainsi fallu recourir à plusieurs versements du budget général pour alimenter le compte cette logique devrait se poursuivre en 2023 alors que les conditions de marché ne sont toujours pas favorables à la réalisation de une nouvelle session les versements du budget général devrait représenter les 3 quarts des recettes du compte et même 95 % une fois les recettes exceptionnelles par ailleurs pour l'année prochaine, seule une faible part des 10 milliards d'euros d'investissement en capital prévues par le gouvernement est connu et détaillée dans le projet annuel de performance du pour 80 % des crédits, le caractère des opérations restent confidentielles, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts patrimoniaux de l'État, si nous pouvons comprendre la question de confidentialité à limite évidemment très fortement la capacité d'appréciation du Parlement pour l'année à venir, par ailleurs, l'inscription de 6,6 milliards d'euros au titre la contribution au désendettement de l'État est un véritable tour de bonneteau budgétaire, selon l'expression de Victorin Lurel dont personne n'est dupe, la contribution au désendettement vient en réalité nourrir d'autant le déficit prévu pour 2023 c'est pour écarter ce mécanisme en trompe-l oeil que la commission des finances, a adopté un amendement visant à supprimer les crédits du programme 732 Ducasse, cet amendement a intervient en cohérence avec l'annulation des crédits proposés sur la mission Engagements financiers de l'État est proposé par notre collègue Jérôme Bascher je tiens cependant à relever un point positif sur le casse le versement sur le cas à la dotation en numéraire du Fonds pour l'innovation de l'industrie J. alors que celle-ci, bénéficier d'une garantie de rémunération de 2,5 % par an sur un compte du Trésor, financé par l'État, le gouvernement faire enfin le choix du bon sens en mettant fin à cette de dotation et en la remplace la remplaçante pardon par des crédits budgétaires, j'en arrive à la situation du portefeuille de l'État actionnaire ce portefeuille de l'État à retrouver cet été une valorisation légèrement supérieur à son niveau d'avant-crise cette valorisation est toutefois dopé par l'homme politique publique d'achat visant les actions d'EDF ainsi si l'on isole la valorisation d'EDF la performance du portefeuille de l'APE est très inférieure à celle des grandes entreprises françaises, et ce malgré les opérations de recopier recapitalisations intervenues la nationalisation d'EDF, il nous semble aller dans le bon sens, elle laisse néanmoins entièrement ouverte la question de la situation financière du groupe, dont la dette devrait atteindre 60 milliards d'euros d'ici la fin de l'année et dans les besoins d'investissement sont évalués entre 17 et 20 milliards d'euros par an, le nouveau président directeur général d'EDF et Luc Rémont qui a pris ses fonctions hier jeudi devra répondre rapidement aux nombreux défis de l'entreprise, il devra rassurer face aux craintes de démantèlement et permettre la viabilité de l'entreprise, je terminerai mon intervention en envisageant la suite quel rôle et quel défi pour l'État actionnaire demain alors que la nouvelle doctrine d'intervention de l'Agence des participations de l'État n'est pas encore défini les pistes esquissées l'an dernier sont toujours le d'actualité : l'intervention de l'APE devrait ainsi ainsi tenir compte 4 facteurs : le soutien auprès d'entreprises touchées par la crise, la préservation de notre souveraineté économique, l'accompagnement des transitions, environnemental et l'accompagnement face aux ruptures technologiques et numériques, outre un retour à la doctrine définie sous François Hollande en 2014, j'y vois surtout le choix de revenir à une utilisation des participations financières de l'État comme un outil de politique économique à part entière, la commission des finances propose donc d'adopter les crédits du compte participation financière de l'État, amendé par l'amendement de la commission visant à supprimer les crédits dédiés aux remboursements factice de la dette, je vous remercie. vous poursuivez Monsieur le Président, puisque maintenant vous maintenant, j'attendais qu'on donne la parole à monsieur Savoldelli

la mission remboursements et dégrèvements retrace les dépenses résultant mécaniquement de l'application de dispositions prévoyant des dégrèvements des remboursements ou des restitutions d'impôts le caractère mécanique de ses dépenses, ces crédits soient évaluatif par ailleurs, cette mission est la première en terme de volume de crédit tous Budgets confondus et permet d'avoir une vision d'ensemble des mesures fiscales mises en oeuvre et de leur évolution, elle se compose de 2 programmes : l'un consacré aux remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, l'autre mêmes opération pour les impôts Directs locaux pour les impôts d'État concernant les remboursements et dégrèvements d'impôts d'État les dépenses soient évalués en PLF à 123,7 milliards d'euros, soit une très légère diminution par rapport à la loi de finances initiale pour 2022 cette quasi-stabilité résulte de tendances contraires entre les différentes actions du programme et je m'attacherai dans le présent à vous à vous faire part des variables les plus notable, tout d'abord les restitutions liée à la mécanique de l'impôt enregistre une hausse importante de 6,6 milliards d'euros entre 2000 22 et 2023 sous l'effet notamment de la hausse des restitutions de TVA qui devrait atteindre en 2023 hein d'otages de 67,2 milliards d'euros, cette augmentation s'explique par le contexte inflationniste en raison de l'effet volume sur la TVA collectée et par le contexte d'incertitude économique qui pousse les entreprises à opter pour le remboursement, plutôt que pour l'imputation du crédit de TVA sur les années suivantes, ce niveau historiquement haut justifierait, à mon sens un renforcement des moyens de lutte contre la fraude à la TVA et une évaluation plus précise des pertes en découlant, ce travail me paraît d'autant plus nécessaire qu'à la suite des différentes réformes de la fiscalité locale, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et baisse des impôts, de production, les collectivités locales bénéficient désormais de fraction de TVA pour un montant total de près de 38 milliards d'euros, ce partage de la TVA entre budget de l'État et collectivités dans le taux de dépendance à cet impôt augmente rend indispensable une gestion optimisée de sa collecte afin de sécuriser les ressources de l'État et des collectivités, maintenant, par ailleurs, en 2023, le niveau des remboursements d'impôt sur les sociétés est évalué à 14,2 milliards d'euros, soit une hausse de 13,8 % par rapport à la LFI 2022 qui résulte d'une diminution attendue du bénéfice fiscal des entreprises en 2022, dans le contexte de crise économique que nous connaissons mais les incertitudes sont grandes sur l'exécution à venir, à l'inverse, et les remboursements liés à des politiques publiques enregistrent une baisse de près de 5 milliards en raison de la suppression du CICE et de la contribution à l'audiovisuel public sur ce point particulier, je m'interroge sur l'effet de cette suppression annoncée comme une mesure pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, ça te suppression ne concernera pas les foyers les plus modestes qui étaient déjà exonérés du paiement de cette contribution, le CIR reste quant à lui stable estimée à environ 7 milliards d'euros en 2023 je demeure sceptique sur l'efficacité de ce dispositif en termes de création d'emplois et de nombre de brevets déposés, comment se satisfaire de l'ambition très mesurée du gouvernement concernant les taux de retour de ce crédit d'impôt avec une cible fixée à un Euro investi pour un euros remboursés, enfin, ce crédit d'impôt est particulièrement complexe à contrôler en raison de la nécessaire coordination entre les services de la DGFIP et ceux du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et génère de nombreux contentieux relatifs au caractère éligible ou non des dépenses d'innovation, il ne faudra donc le réformer je conclurai c'était parti sur les remboursements d'impôts d'État par une note positive, les remboursements liés au contentieux de série baisse sensiblement en raison des efforts notables faits dans le suivi des plus gros contentieux pour les impôts locaux, je suis tout être pendant quelques instants en PLF 2023 les crédits évalués au titre 200 hein s'élève à 4,6 milliards d'euros, soit une baisse de 30,8 % par rapport à la LFI 2022 cette diminution fait suite aux baisses consécutives enregistrées lors des précédents elle qui s'explique notamment par la réforme ta taxe d'habitation sur les résidences principales et dans une moindre pot portions par la réforme des impôts, de production et comme Savoldelli m'a donné un document, un peu long, je vais être obligé de le réduire en disant qu'il ne faudrait pas rendre encore plus illisible, le financement des collectivités locales, territoriales, au final, les mesures de compensation des différentes réformes de la fiscalité locale génère une perte de l'autonomie financière des collectivités territoriales en 2022, la part de TVA et déjà la première recettes des départements et des régions après la possible suppression de la CVAE, elle deviendra la 2ème du bloc communal ainsi les ressources et l'avenir des collectivités vont 2 heures mais être tributaire en majorité d'un impôt national sur lequel elle n'exerce aucun pouvoir de taux et la dynamique importante certes, dans cette période inflationniste mais dont les évolutions futures reste très incertaine.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous prie d'excuser Martine Berthet, qui m'a chargé de la remplacer la commission des affaires économiques, a émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de ce compte, la compétence et le travail du personnel de l'Agence des participations de l'État ne sont bien évidemment pas en cause, mais nous regrettons et contestant les faiblesses du gouvernement en ce qui concerne l'État actionnaire, la première raison, et le fait qu'en dépit d'annonces qui allait dans le bon sens, le gouvernement n'a toujours pas fait le choix d'opter pour un État stratège capable de soutenir résolument la souveraineté économique de la France, la défense de cette dernière, elle reste balbutiante et la nationalisation d'EDF ne doit pas nous tromper, elle est l'arbre qui cache une forêt d'internautes notamment de renoncement et d'hésitations, en effet, nous avons toujours considéré que la doctrine d'investissement formulées en 2017 étaient trop flou et ne garantissait pas en l'état, la sauvegarde de la souveraineté économique française l'enchaînement de crise depuis 2020, a mis sur le devant de la scène nombres de produits entreprises aux filières qui seront stratégique pour notre pays et qui pour autant ne rentre pas dans les catégories que vous aviez défini l'an dernier, nous avons donc accueilli avec satisfaction les propos du ministre et du commissaire aux participations selon lesquelles l'État actionnaire aller davantage prendre en compte cette dimension de souveraineté, c'est-à-dire exactement ce que nous martelant au Sénat depuis des années, malheureusement, 3 ans après le début de la crise, nous devons toujours attendent de la traduction concrète de ces déclarations, alors même que la nouvelle doctrine n'est toujours pas publié par ailleurs en ce qui concerne la nationalisation d'EDF, nous n'en savons pas beaucoup plus que ce que nous avons pu lire dans la presse, les informations utiles sont assez rares en dépit du montant important de l'opération. Et la nationalisation ne répond pas à toutes les questions, par exemple, comment régler la dette de près de 43 milliards d'euros d'EDF, comment sera financée la relance du nucléaire qu'on est-il des contentieux relatif aux concessions hydrauliques, nous regrettons également fortement la méthode par laquelle le gouvernement envisage de se désendetter de 7 milliards d'euros grâce à ce compte, alors même qu'il ne prévoit aucune recette pour le le dire autrement, le remboursement de la dette proviendra en réalité d'un simple versement du budget général, le tour de passe-passe est vertigineux en prend 7 milliards dans le budget, on les met dans le conte qui nous intéresse et on les verse au désendettement, autrement dit, il n'y a absolument aucun effort structurel qui est fait pour assainir les finances publiques. On ne rembourse pas la dette par des économies, mais en continuant de creuser le budget général tout cela simplement pour afficher un effort de danse désendettement mais qui n'en n'a que le nom, car cela revient en fait à s'endetter pour se désendetter, voilà, mes chers collègues, 3 raisons qui conduisent la Commission a donné un avis défavorable à l'approbation de ce compte. Je vous remercie,

l'objet de ces biches, on ne peut paraître quelque peu aride, il n'en est moi point crucial d'abord par les masses financières qui les représentent les engagements financiers de l'État, cette plus de 50 milliards d'euros et les remboursements gravement plus de 120 milliards d'euros, sans compter les différents comptes spéciaux, le budget de la mission Engagements financiers augmentent de plus de 35 % en fait de paiement en 2023, le montant total représenterait plus de 10 % des dépenses de l'État la caractère en de cette mission, c'est l'augmentation de la charge de la dette, la remontée des taux d'intérêt depuis le début de 2022, a eu un effet quasi immédiat sur le coup de l'entrée de la demande publique qui était resté somme toute limité ces dernières années malgré un encours total qui a littéralement explosé d'abord après la crise financière de les 3 années qui ont suivi, mais surtout en 2020, 2021, avec les mesures liées à la crise sanitaire, plus que jamais notre État vit à crédit pouvant encore compter sur la qualité de la signature française sur les marchés internationaux, la remontée pour ta spectaculaire : près de 12 milliards d'euros supplémentaires pour le seul paiement des intérêts d'emprunt dès cette année par rapport à la loi de fédérer initial en 2023, le service de la théâtre de 24 à peu près équivalent à 50 d'euros il dépassera de nouveau le budget de la Défense réalité quelque peu ironique alors au un sens de l'effort militaire face à la nouvelle donne internationale face au durcissement du marché obligataire, l'Agence France Trésor n'aura pas intérêt à rechercher davantage les faveurs d'investisseurs français plutôt qu'internationaux afin de réduire les risques de s'ouvre noter de notre dette publique, à l'instar du Japon qui connaît la date public le plus élevé du monde, mais essentiellement détenu par des résidents, il est vrai que cela ne colle pas trop avec les concessions hors libérale qui prévalent au sein de la zone Euro, sur l'imputation de la dette Covid dans un programme budgétaire dédiée j'émettrai n'même réserve que la commission des finances, d'abord sur les modalités de calcul à la suite sur le principe même, l'argument de la meilleure éligibilité ne pas faire oublier que les mêmes règles s'appliquent à ce qui concerne le remboursement du capital et le paiement des intérêts, l'ensemble des dates public est intégré dans la fameuse date Maastricht étalon commun aux pays européens et instrument de mesure de la Commission de Bruxelles, les montants énormes de la mission remboursements elle gravement de son jardin Roman décompté dans la presse à de la présentation courante courant de du budget de l'État, il est vrai qu'il y a semble-t-il peu à développer sur cette mission s'agissant de restitution d'impôts et taxes par l'administration fiscale, la taille du montant interroge néanmoins sur l'ampleur des irrégularités dans la perception des impôts, mais encore une fois, et il s'agit davantage donne débat de spécialistes du cours recouvrement fiscal de dégrèvements d'impôts sont plus aspirant sa suppression de la part régionale aussi eux cette année et la suppression générale prévue pour 2023 et 2024 de 24 comme ici à l'euro près ou bien le dégrèvement de 50 % aux entreprises si le si si le vote du Sénat venait à être définitivement retenu donnerait lieu automatiquement à une hausse significative des mouvements sur ce compte, en conclusion, et malgré ces réserves, le groupe RDSE approuvera les crédits de cette nuit. Merci Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au tournant du siècle, la France s'est laissé bercer par le mythe d'une mondialisation heureuse cette douce musique nous a fait oublier l'importance de l'État, stratège malheureusement la crise sanitaire, d'abord, puis la crise énergétique nous ont cruellement rappelé sa nécessité, l'État, stratège, c'est l'État qui bâtit une stratégie économique pour défendre sa souveraineté, il ne s'agit pas de dire que l'État doit, a dit le ministre et l'économie, bien au contraire, l'État doit choisir ses priorités stratégiques et travailler sur ces à garantir l'intérêt général sur le long terme, c'est cette vision de l'État, stratège qui doit aujourd'hui nous réunir au-delà de nos clivages politiques, vous l'aurez compris je concentrerai mon propos sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État, ce compte a vu ses crédits augmenter depuis le début de la crise sanitaire, il y a près de 3 ans, cela correspond précisément au retour de l'État, stratège sur le devant de la scène en 2023 les crédits dépasseront les 17 milliards d'euros, essentiellement en provenance du budget général, la succession des crises, a eu un double effet positif d'une part, elle a permis l'abondement massif de ce compte pour financer une stratégie économique ambitieuse, d'autre part, elle a encouragé l'Agence des participations de l'État à à reconsidérer sa doctrine pour se consacrer désormais sur les secteurs les plus stratégiques, c'est le cas avec la nationalisation d'EDF cette nationalisation prépare le renouvellement de notre parc nucléaire, avec la construction de réacteurs EPR à long terme, en cohérence avec la volonté affichée par le gouvernement de neutralité carbone et d'indépendance énergétique, bien sûr, l'avenir d'EDF ne tient pas exclusivement à ces nouveaux chantiers notre fleuron national devra également rénover le parc existant, développe des produits d'export tels que Les SMR, hé bien sûr poursuivre le développement des énergies renouvelables, afin de doter la France de mix des Camerounais Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui nous tiennent depuis longtemps à coeur, c'est notamment le renouvellement des concessions électrique, nous avons en Aveyron, cela fait 10 ans que c'est le six, sont en cours et suspendu à la décision de la Commission européenne et c'est le gouvernement qui doit négocier avec elle, nous souhaitons quand j'étais déjà député et encore aujourd'hui, les sénateurs, me semble-t-il, l'ensemble de des formations politiques qu'EDF continue à avoir ce là pourquoi parce qu'il EDF a envie de considérablement investir sur ses barrages hydroélectriques et sachez qu'un navire en ils représentent 10 % de la production hydroélectrique national et on sait combien aujourd'hui, c'est le s'il est nécessaire et en quelques secondes, on peut offrir aux réseaux une quantité considérablement d'énergie, je crois que ce n'est pas neutre dans cette, dans cette période, donc nous aimerions que ce dossier avance, je crois que pour toutes ces missions, la nationalisation d'EDF contribuera à atteindre ses objectifs, je tiens ici à saluer le travail mené par notre collègue Martine Berthet, rapporteur spécial au nom de la commission des affaires économiques sur ces crédits, je partage l'essentiel de son analyse, notamment concernant les enjeux liés à la nationalisation d'EDF et au grand professionnalisme de l'Agence des participations de l'État, je partage également ses réserves quant à la la lisibilité du compte des montants importants sont transférés du budget général vers ce compte spécial, ce qui permet de soutenir une politique ambitieuse, mais ce qu'il doit aussi s'accompagner de décision courageuse, d'autre part, la nouvelle doctrine de l'agence doit également permettre la cession d'actifs non stratégiques pour poursuivre le désendettement de l'État, malgré ces réserves, notre groupe les indépendants souhaite soutenir les crédits de ce compte spécial il ne si j'ai, il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au gouvernement, mais bien de renforcer le rôle de l'État, stratège dans notre pays. Merci. Et la parole est maintenant monsieur Daniel Breuiller pour le groupe Écologie Solidarité territoire et pour quatre minutes. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, monsieur le Ministre, chers collègues, il faut arrêter de confier à Jérôme Bascher, la mission chaque fois qu'il la présente la dette augmente. La mission Engagements financiers de l'État est en hausse, dit-il, et il pointe à raison que c'est dû à un double effet : un effet taux un effet volume plusieurs composantes dans l'effet volume une dette Covid conséquence du du quoi qu'il en coûte, dans une période où ceux qui prône l'orthodoxie budgétaire, c'était justement converti à la nécessaire intervention massive de l'État, un déficit de l'État au nom duquel le gouvernement impose ou voudrait imposer des restrictions budgétaires aux collectivités locales, des mesures de soutien face à l'inflation, alors quand les taux repartent à la hausse, la charge de la dette augmente de 50 milliards mais ces sommes ne sont pas perdus pour tout le monde, car si l'État est endetté, il y a en face des prêteurs dont les profits vont augmenter au même rythme, profitant de l'inflation, encore une fois, je le dis face aux crises face aux crises à venir face aux crises climatiques dont les coûts seront sans aucune mesure avec les coûts déjà trop élevé de l'été catastrophique que nous venons de vivre, nous devons nous interroger sur notre manière de gérer la dette la dette Covid est isolé et si monsieur le rapporteur spécial estime à juste titre qu'il n'y a aucun argument économique ou budgétaire pour justifier cet isolement, nous pensons qu'il y en a un pour isoler, en revanche, la dette liée aux mesures environnementales parce qu'elle n'a pas la même nature parce que la noyé dans la masse indistincte de la dette va conduire une fois encore à la traiter comme une variable d'ajustement et le gouvernement va encore nous proposer son arbitrage : d'abord on maîtrise la dette, ensuite on prend les mesures nécessaires pour s'engager plus radicalement contre le réchauffement climatique pour s'en donner les moyens, ne faut-il pas, je le répète à nouveau, Monsieur le Ministre, stopper le désarmement fiscal de l'État d'imiter l'effet volume avec la mise en place de recettes nouvelles, comme par exemple l'ISF climatique dont j'espère que vous avez lu l'intégralité de notre proposition concernant la mission remboursements et dégrèvements, nous nous prononçons sur des crédits qui, en raison du caractère mécanique de ces dépenses sont évaluatif comme l'a noté le rapporteur spécial Pascal Savoldelli sous la voix du président rénale cependant ces prévisions peuvent susciter quelques interrogations, l'impôt sur les sociétés en 2023, le rapport indique que le niveau estimé des remboursements d'impôts est en hausse de 13,8 par rapport à la et les filles 2022 ces remboursements correspondent à l'écart entre l'imposition effectivement du et les acomptes calculés sur les résultats de l'année précédente, cette augmentation de remboursement et donc liée à la baisse attendue du bénéfice fiscal des entreprises en 2022, dans un contexte de crise inflationniste, j'ai quelques difficultés à rapprocher cette information baisse attendue du bénéfice fiscal des entreprises dans un contexte de crise inflationniste à votre déclaration de Monsieur le Ministre, dans l'hémicycle 21 novembre plus gâteau grandit, plus les recettes fiscales augmentent, nous percevons davantage d'impôt sur les sociétés, depuis que le taux a été abaissé à 25 % sur la question récurrente de la fraude à la TVA, la nécessité d'une vigilance accrue sur les risques de montages frauduleux et pointé et nous soutenons toutes les mesures prises, qui nécessitent, selon nous, une hausse des moyens humains qui, par ailleurs, génère des recettes bien supérieur au coût des postes qui sont consacrés. Si la parole est maintenant Monsieur Thani Mohamed Soihili et ce pour quatre minutes pour le groupe du Rassemblement démocratique progressiste et indépendant. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances Madame messieurs les rapporteurs spéciaux plein de relance, France 2000 Trent bouclier tarifaire, le gouvernement a fait ce choix volontariste qui consiste à soutenir coûte que coûte, notre économie, considérant que cet accompagnement pour recréer de la richesse, si je rappelle ici le quoi qu'il en coûte, c'est que ce plan de soutien, a eu un impact sur nos comptes publics de 5 milliards d'euros, ce n'est pas rien, mais c'est une stratégie pleinement assumé qui a permis de sauver notre économie, de fait, les crédits de la mission Engagements financiers de l'État affiche une hausse inédite de 15 9 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2022 il s'établirait ainsi à 60 virgule 2 milliards d'euros en 2023, cette augmentation s'explique principalement par l'ouverture, un cours d'année de 11,9 milliards d'euros supplémentaires pour financer la charge de la dette dans un contexte de forte inflation, la maîtrise de l'inflation en France contribue toutefois à modérer ce facteur en parallèle cette même inflation élevée a également conduit les banques centrales à normaliser leurs politiques monétaire et à remonter leurs taux d'intérêt après plusieurs années de conditions extrêmement favorables pour le financement de la dette française, les taux d'intérêt augmenteraient significativement en 2023 à 2,6 % en moyenne annuelle pour les obligations assimilables du Trésor à 10 ans, c'est donc la fin de l'argent magique, c'est-à-dire la fin de l'assouplissement quantitatif prônée par la BCE, qui avait été abondamment utilisé durant la décennie 2010 aussi face au spectre de la dette et pour éviter de remontrances du FMI notre gouvernement ne regarde pas ailleurs, c'est pour cela que le quoi qu'il en coûte, se mue à combien ça coûte, c'est aussi pour cela que nous sommes convaincus que les réformes structurelles, comme le recul de l'âge du départ à la retraite ou l'achèvement de la réforme de l'assurance chômage sont des réformes nécessaires qui conduiront à échéance à la maîtrise de nos dépenses publiques, c'est un ce sens que le programme 114 relatifs aux prêts garantis par l'État va poursuivre sa décrue, la mobilisation toujours forte de cette action de l'ordre de 1,91 milliards d'euros, baisse de 30 % par rapport à 2022, rappelons-nous, dans le sillage du quoi qu'il a un coût : le prix garanti par l'État, avait connu un grand succès au 31 juillet 2022, on dénombrait près de 800000 entreprises bénéficiaires du PGE pour un concours total de 142 virgule 7 milliards d'euros, mais l'heure est désormais aux remboursements, selon le dernier baromètre des pays France, publiée ce jeudi 9 % des PME, TPE et 1 souscrit au PGE redoutent de ne pas être en mesure de rembourser la proportion est en hausse de 2 points par rapport à la dernière enquête en date, mais dans leur grande majorité, les entreprises devraient honorer leurs échéances, par ailleurs, le compte d'affectation spéciale relatif au principal oh participation financière de l'État, la nationalisation d'EDF constitue en effet une étape indispensable pour renforcer la crédibilité de l'entreprise par les marchés face au programme de construction de Six EPR pour poursuivre le programme du grand carénage et pour amplifier les investissements dans les énergies renouvelables sur la mission remboursements et dégrèvements il faut notamment il faut noter que les remboursements d'impôts d'État lié au contentieux de série baisse sensiblement, passant ainsi de 2,7 milliards en 2022 à 1 virgule 1 milliard d'euros en raison des efforts réalisés dans le suivi des plus gros contentieux, nous ne pouvons que saluer ici le travers ne travail réalisé par notre administration fiscale pour conclure, nous pourrions représenté la France sur une ligne de crête pris un étau entre le rétablissement nécessaire de nos comptes publics et le soutien de notre activité économique et énergétique, c'est toutefois ce ce chemin que nous devons poursuivre.

Madame la présidente, monsieur le ministre à monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, la mission Engagements financiers de l'État, appellent à une grande vigilance de notre part en raison de nombreuses zones d'ombre autour de ces programmes ainsi plusieurs points méritent notre attention, tout d'abord, la charge de la dette, a littéralement explosé entre 2020 et 2 A et 2023 en passant à 45, les crédits de la mission sont parmi ceux qui augmente le plus en raison de cette inflation constante que nous subissons depuis maintenant quelques mois face à une hausse historique des taux d'intérêt, on peut légitimement s'interroger sur vos prévisions de stabilité à l'horizon 2023, ensuite les prêts garantis par l'État, PGE risque fort d'être une véritable bombe à retardement en effet la crise sanitaire, les conséquences économiques de la crise en Ukraine, crise de l'énergie ou de l'approvisionnement, coût des matières premières les tensions sur le marché du travail ont eu de fortes répercussions sur la trésorerie des entreprises le risque ici est double : d'une part, une accélération du nombre de faillites, y compris d'entreprise parfaitement viable et productive, et, d'autre part une réduction de leurs dépenses d'investissement. Il s'agit là de ce que les économistes qualifient généralement d'étranglement par la dette et les chiffres sont édifiants : près de 700000 entreprises ont souscrit un PGE pour plus de 148 milliards d'euros au total, seule, hein, pour 100 d'entre elles se sont aujourd'hui acquittés de leurs dettes,

bien que le PLFR 2022 prévoit une baisse de 2 milliards d'euros des provisions pour les prêts garantis par l'État, nous avons de sérieux doutes sur ce calibrage en 2023 tout comme nous pensons qu'il est urgent de mettre en place des mécanismes innovants pour éviter le défaut de paiement des créances aux entreprises dont la solvabilité à court terme est remise en question, enfin, que penser de l'absence de prise en compte budgétaires de la dette Covid ou de la dette de SNCF, réseau parmi les crédits dévolus à la charge de la dette, alors qu'en toute logique, ce devrait être, ce aussi au regard de toutes ces approximations se pose encore plus aujourd'hui, là, la question du désarmement fiscal de la France, l'amortissement de ses dettes, doit-il se faire sur le dos de tous les Français, en tablant sur une réduction de la dépense publique et en supprimant encore plus de service public, nous ne le pensons pas, bien au contraire, nous avons formulé des propositions pour davantage de justice fiscale et sociale, en revenant sur la question de la flotte taxe le rétablissement de l'ISF : la taxation des superprofits le rehaussement de la taxe sur le numérique, manifestement, les débats sur la première partie de ce PLF pour 2023 n'indique aucune remise en question de vos choix fiscaux, vous refusez toujours de faire payer ceux qui le peuvent, les plus aisés, ceux qui s'enrichissent de la crise et de la situation économique du pays au détriment des plus vulnérables, Ministre, fragilise la situation financière de notre pays et participe à ce sentiment d'injustice et d'abandon qui gagne un peu plus chaque jour l'ensemble de nos concitoyens, cette fracture se manifeste dans l'accès aux services publics, car les démettre dématérialisation est aussi une facilité qui isole et cela même si ça semble être le cas si je rappelle que la dématérialisation ne peut se substituer à l'accueil du public, pour qui la fracture numérique est un handicap de tous les jours, enfin l'analyse du programme 200 remboursements et dégrèvements d'impôts locaux amène tout de même à quelques commentaires en volume, nous constatons une baisse de 31 % environ par rapport à l'exercice précédent, cette baisse continue n'est pas une simple ligne comptable, elle traduit de manière indirecte, l'insidieuse atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités en effet cette diminution découle de la suppression progressive de la taxe d'habitation, d'une part et de la réduction massive des impôts, de production, vous le savez, Monsieur le Ministre, nous sommes loin de partager votre position dogmatique de la baisse d'impôts qui conduit à une injustice grandissante d'ailleurs au rythme où vont les où vont vos réformes, il est à craindre de ne plus avoir à étudié ce programme l'an prochain car sans impôts locaux, point de remboursement ou de dégrèvement

certains programmes budgétaires pourraient disparaître et avec eux, une certaine idée de la décentralisation, je vous remercie. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, excusez mon collègue Fabien Gay en raison des changements d'ordre du jour sous ces dernières 24 heures à travers la discussion du compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État, qui retrace la doctrine de l'État actionnaire, je souhaite particulièrement insisté sur l'avenir du groupe EDF, en effet, après une augmentation de 2 6 milliards d'euros en avril 2022 justifiée par la situation financière très difficile de l'entreprise, à noter que cette situation est due aussi aux contraintes que l'État a imposé à EDF, déblocage de prix des tarifs de l'électricité, les crédits doivent désormais être employé pour financer la montée au capital du groupe EDF pour parvenir à 100 pour 100 de détention par l'État ont rachetant les parts des actionnaires minoritaires, alors que cette opération a un coût annoncé de 9 7 milliards d'euros, le Parlement ne dispose pas d'informations précises sur les raisons d'une telle opération ni sur votre vision stratégique pour la suite de l'entreprise historique, les documents budgétaires en notre possession sont incomplets, voire inexistants et vous refusez toujours au débat, pourquoi, de plus, de nombreuses interrogations voire zones d'ombres persistent, hormis la volonté d'afficher afficher de gérer les concessions hydroélectriques en quasi-régie afin d'éviter leur mise en concurrence, qu'attendez-vous d'une détention de 5 % du capital d'EDF, avez-vous abandonné la réorganisation groupe EDF sur le modèle du projet Hercule ou grand EDF impliquant le démantèlement de l'entreprise et la privatisation de ses activités les plus rentables, en particulier les énergies renouvelables, sur ce dernier point, pourquoi les notes préparatoires à l'opération montée au capital qui indiquerait qu'elle permettrait de préparer sur une base nouvelle, les négociations régulation du nucléaire et réorganisation du groupe à venir avec l'ensemble des parties prenantes ne sont toujours pas accessibles aux parlementaires allez-vous céder des actifs comme Dalkia ouvrir au capital enedis dois-je rappeler qu'EDF est au coeur de notre système électrique, dès lors, il est impératif qu'il y ait le plus de transparence possible quant au futur statut du groupe du devenir du mécanisme à Rennes et du financement du nouveau nucléaire qui seront les grands sujets de l'un de l'année à venir face aux enjeux financiers de cette montée au capital en pleine crise énergétique et d'approvisionnement, le gouvernement ne peut faire l'économie d'une explication devant le Parlement, comme cela a été rappelé sur de nombreux bancs dans notre hémicycle l'absence de recours à une loi de nationalisation ne permet pas d'avoir un débat satisfaisant sur l'avenir de l'entreprise sur l'emploi des deniers publics nécessaires pour mener à bien cette étatisation parce qu'EDF est une entreprise stratégique, contribuant à la souveraineté énergétique du pays, Pascal en charge une mission d'intérêt général et de service public, nous pensons que sa disparition dans sa forme intégré porte en elle le germe d'un risque systématique comme vous le savez, nous sommes favorables à une nationalisation d'EDF nous sommes favorables à la reconstruction d'un grand service public de l'énergie qui regrouperait NJ et pourquoi pas à Total un service public de l'énergie soustrait aux logique concurrentielle du marché européen, c'est pourquoi notre groupe rejettera les crédits de ce compte, nous voulons rappeler au gouvernement la nécessité d'avoir un tel débat sur la stratégie d'EDF, le débat doit concerner le Parlement en associant aussi les usagers, les salariés et les syndicats du groupe, je vous remercie. Merci madame Goulet pour 6 minutes pour le groupe Union centriste. La présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, avec Laurent Saint-Martin il y a quelques années nous avions envisagé d'avoir un débat sur la dette avant tout début du PLF parce qu'en réalité le déficit et la dette Anil un peu notre. Entre liberté et je pense que ce débat extrêmement important, je rejoindrai les propos du rapporteur sur une mission que j'affectionne particulièrement, puisque j'étais moi-même rapporteur de cette mission, quand j'ai eu le bonheur de siéger à la commission des finances pendant 3 ans. Donc je vois bien de quoi il s'agit et et notamment les effets anesthésiants ces dernières années d'un taux négatif de Qui évidemment anesthésiée complètement la moindre, la moindre réaction et on n'a pas arrêté de dire mais un beau jour, comme la Belle au bois dormant, il va falloir se réveiller les taux vont augmenter, ça va arriver, mais telle soeur Anne, ne vois rien venir, évidemment, personne ne s'inquiéter de l'augmentation des taux qui allait venir puisqu'il arrivait pas cette fois-ci c'est fait, et donc nous voilà avec un réveil difficile je voudrais donc évidemment félicité. Es le rapporteur pour cette mission et aussi vous dire, Monsieur le Ministre, qu'à plusieurs reprises il y a donc quelques années, on avait envie d'une on avait demandé une simulation des conséquences d'une augmentation des taux et chacun des interlocuteurs qu'on avait au moment des auditions se renvoyer la patate chaude en disant nous on sait pas faire ses simulations, on ne peut pas le faire, et le vrai, de l'augmentation des taux, mais je pense que si par hasard ça continuer comme ça, ce serait quand même assez intéressant de pouvoir avoir des des évaluations des conséquences immédiates de l'augmentation des taux. Au moins pour pour l'année prochaine je voudrais à ce à ce moment précis, saluer les agents de France Trésor, qui font quand même un travail absolument remarquable dans des conditions pas forcément facile et vous demander, monsieur le ministre, si vous pouviez avoir la liste des possesseurs de notre dette et comment comment elle est répartie, ce serait aussi intéressant à avoir puisqu'on a un certain nombre de données, mais pas forcément toutes les données à partir du moment où ce sujet devient tellement fragile, sachant que nous avons aussi et ça va être le le propos majeur que je vais développer maintenant qui est le problème des engagements hors bilan les, les, les engagements hors bilan c'est 4615 milliards d'euros, c'est quand même pas complètement rien nous avons sur ce sujet des interrogations certaines donc je ne sais pas si vous pourrez nous donner quelques informations sur ce sujet, sachant que, à cette heure tardive, la façon d'être populaire dans cette maison, c'est de parler 3 minutes au lieu de 6.

de l'Orne, voilà et je voudrais à ce moment, remercier les membres de la commission des lois qui sont majoritairement présents sur ce sujet important sans plaisanterie, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, je crois qu'il faudrait essayer l'année prochaine que ce débat figure assez tôt dans l'ordre du jour parce qu'il arrive toujours le tard le soir, c'est un débat, sacrifié, alors que, à mon sens, c'est un débat absolument fondamental pour la compréhension de l'équilibre budgétaire et aussi des moyens dont on dispose pour les politiques publiques, donc au au delà du caractère mécanique de la reprise du rapport du rapporteur c'est un c'est un dossier extrêmement important comme le dossier d'ailleurs des dégrèvements est un dossier les dégrèvements les dégrèvements, c'est une politique, c'est une stratégie et donc je trouve extrêmement dommageable que cette année comme l'année d'avant l'année d'avant et l'année encore d'avant ce débat arrive à cette heure tardive, je crois que c'est un débat très important. Et je continue à penser que ce ce dont on avait parlé à l'époque avec le député Saint- Martin s'applique encore cette année et qu'il faudrait peut-être l'année prochaine en début de session budgétaire à voir monsieur le président de la commission des finances, un débat uniquement sur les engagements et donc sur la dette, de façon à ce qu'on soit totalement éclairé sur les disponibilités qu'on pourrait avoir sur les politiques publiques à venir, je vous remercie de votre attention.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs, mesdames, messieurs les rapporteurs spéciaux, rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier les rapporteurs et les orateurs des groupes pour la qualité de leurs interventions et je m'efforcerai dans le temps imparti de répondre aux principaux sujets soulevés et mon propos autour des 3 blocs de politique publique examiné dans cette discussion, d'abord, concernant les engagements financiers de l'État, je veux dire que nous partageons bien évidemment la préoccupation exprimée par le rapporteur, Jérôme Bascher et plusieurs d'entre vous, sur l'évolution des taux d'intérêt, la programmation budgétaire du gouvernement intègre déjà une hausse des taux d'intérêt en cohérence avec un scénario pluriannuelle de normalisation des conditions monétaires, le scénario de taux retenu pour le projet de loi de finances et celui d'une remontée des taux longs ainsi le projet de loi de finances fait l'hypothèse que le taux à 10 ans serait à 2 5 % fin 2022 puis à 2 6 % fin 2023, j'ai entendu monsieur Villach qui a posé la question de ses taux, non pardon, c'était Madame Briquet qui a posé la question des ses prévisions de taux et qui a remis en question, en tout cas, interrogé nos prévisions de de 6 à fin 2023 ce soir, l'OAT à 10 ans, état de 43 la prévision des marchés pour la fin 2022 est égal ou inférieur à 2,5 % et le budget 2023 est bâti sur des hypothèses structurelle et non sur les dernières données du marché qui est évidemment très volatile en ce moment, j'en profite et je fais une hantise pour répondre à monsieur qui a posé la question en tout cas qu'il a dit souhaiter que à l'Agence France Trésor reviennent sur son marché domestique, je veux dire que la diversité, la diversité des investisseurs internationaux est un atout et non une menace, ça nous permet d'emprunter moins cher, ça nous permet de diversifier les détenteurs et de les mettre en concurrence et je veux rappeler que détenir une OAT n'ouvre qu'un seul droit, celui d'être remboursé je viens ensuite sur la question Madame Goulet sur les prévisions d'pacte d'une augmentation des taux, un choc de taux de 1 point par rapport au scénario de référence qui est à deux 6 entraînerait plus de 5 milliards la première année, 6 milliards la deuxième année et 16 milliards à horizon 2027, on voit donc l'enjeu absolument majeur sur ce sujet, le scénario de hausse progressive des taux d'intérêt d'ailleurs est cohérent avec le scénario macroéconomique du gouvernement, ce scénario est également cohérent avec la cible d'inflation à long terme de la Banque centrale européenne dont le mandat est de maintenir l'inflation, l'inflation de long terme, proche de 2 je souhaite rappeler ensuite que le calibrage d'un montant retenu pour les appels en garantie, qui a été critiquée par Madame Briquet en 2023 des prêts garantis par l'État prend appui sur les calculs réalisés par la Banque de France pour la DG Trésor et actualisé au moins 2 fois par an, l'évolution des appels en garantie dépend étroitement de l'évolution de la conjoncture économique et financière de la dynamique des défaillances d'entreprises et de la bonne santé financière des entreprises, je pense au prix des intrants aux coûts de production à l'accès au financement liquidités au niveau d'endettement, c'est pourquoi aucun autre élément que les prévisions susmentionnées ne permet de présager d'un montant final d'avances sur indemnisation pour l'année 2000 23 au sujet de la dette Covid enfin l'isolement budgétaire qui a été relevé, ce n'est critiqué par messieurs Bachere et rénale dans un programme dédié à pour objectif prioritaire de retracer dans les comptes publics de manière lisible et clair, le montant de dettes d'État résultant de la crise sanitaire et d'afficher une trajectoire de remboursement de cette dette entre 2000 22 et 2042 l'intégration de la charge des intérêts avec la dette elles-mêmes qui matérialise le coût complet de l'effort national est effectivement inhabituel mais s'apprécie au regard de sa vertu pédagogique je suis les participation financière de l'État, pour commencer, je rappelle que, de manière constante, tous les gouvernements ont fait le choix de retenir un montant notionnel de prévisions de recettes et de dépenses afin de ne pas donner de signaux aux marchés, le gouvernement est en effet soumis à plusieurs obligations celle évidemment la première de l'information et de la transparence à l'égard du Parlement, celle de gérer au mieux les données publiques et donc de défendre les intérêts du contribuable, ce qui suppose de ne pas révéler ses intentions au marché celle de protéger la réputation d'entreprise dont les difficultés potentielles pourraient nécessiter en cours d'année, des opérations de recapitalisation, c'est cette tension entre ces impératifs qui s'imposent au gouvernement qui justifie cette inscription de crédits notionnel soulignée par Madame Michèle Jacques dans son intervention, malgré ces contraintes, l'effort de transparence de l'État et chaque année particulièrement important avec la publication en annexe du PLF du projet annuel de performance du compte d'affectation spéciale ainsi que d'un rapport d'activité dans rapport financier de l'Agence des participations de l'État, en réponse à Madame Jacques notre vision d'un état stratège existe bel et bien elle se concrétise en recourant à 3 outils d'intervention en fonds propres et dont les doctrines sont complémentaires la Caisse des dépôts et consignations investissent sans horizon de temps en tant qu'actionnaire stratégique d'influence ou de contrôle dans certains secteurs prioritaires, je pense évidemment à la transition écologique au développement économique à la cohésion territoriale à l'habitat, la cohésion sociale, mais elle reste évidemment également attaché à des niveaux de rentabilité minimum la BPI en tant qu'actionnaire minoritaire actif au capital d'entreprises françaises, à l'occasion d'une évolution actionnariale et aux côtés d'un actionnaire majoritaire ou de référence pour assurer un actionnariat français dans ces entreprises avec un horizon d'investissement de type fonds d'investissement, même si la durée de détention n'est pas fixé exemptés l'APE est pour sa part l'actionnaire stratégique sur les sujets les plus critiques, conjuguant un fort niveau de contrôle de l'État 44 entreprises dans lesquelles l'État est majoritaire sur 83, une capacité à privilégier des objectifs stratégiques ou industriels avant les attentes de rendement et des capacités financières pouvant être gérés sur le long terme et sans limite d'horizon d'investissement, c'est dans ce contexte que doit s'apprécier la performance financière du portefeuille coté de l'APE ce portefeuille est fortement pondéré sur un petit nombre de secteurs, dont celui de l'énergie, ce qui limite sa comparabilité avec le panel plus large des entreprises du CAC 40 évidemment au 18 novembre 2022, la valeur des participations de l'État dans EDF et Engie ainsi, 56 % de la valeur du portefeuille côté État pour terminer je souhaite répondre à la question soulevée régulièrement sur l'inscription de 6 6 milliards d'euros au titre de la contribution au désendettement de l'État, nous avons mis en place une trajectoire d'apurement de la dette née de la crise sanitaire permettant d'amortir sur une période de 20 ans, le montant de la dette Covid par des dotations annuelles auprès de la Caisse de la dette publique, en l'absence de recettes de cession et compte tenu du caractère stratégique de la dépense, chaque échéance annuelle versée à la CDP nécessite l'abondement préalables en recettes du CAS PFE à partir du programme 369 c'est-à-dire le programme amortissement de la dette liée à la Covid 19 à hauteur de la dépense envisagée : maintenir la maquette budgétaire inchangé, je le dis en conservant le programme 732 permettra d'assurer le suivi dans le temps de ces opérations, notamment quand une reprise des cessions de participations pourra être envisagée pour participer au désendettement, c'est notre souhait, ensuite concernant les remboursements et dégrèvements en 1er lieu la hausse marquée du remboursement de la TVA traduit une préférence pour le présent de la part des entreprises dans un contexte d'incertitude économique en ce qu'ils contribuent à la liquidité des entreprises le droit d'opter pour le remboursement, plutôt pour l'imputation pour les périodes d'affaire suivante participe donc très concrètement au soutien de l'économie, c'est un outil qui a été mobilisés de façon très efficace dans les premiers mois de la crise sanitaire, il fait partie des aides peu visible mais décisive pour nos entreprises, s'agissant des principes fiscaux, je vous rappelle que la TVA est censé rester neutre pour les acteurs économiques, tout au long de la chaîne de valeur et que la charge de trésorerie lié au décalage entre la collecte et le reversement de la TVA peu représenter dans certains secteurs et en période de tensions économiques une charge réelle pour les exploitations, ce dispositif de remboursement de TVA constituent une part majoritaire des crédits de la mission c'est en parallèle je veux indiquer que la lutte contre la fraude à la TVA et l'un des objectifs prioritaires du gouvernement et c'est un domaine dans lequel nous ne ménageons pas nos efforts, je regarde évidemment Madame Goulet, spécialiste de la fraude en 1er lieu les travaux d'estimation du manque à gagner en matière de TVA progressent avec la mise au point par l'Insee d'une méthode d'évaluation robuste, nous les premiers résultats donnent une enveloppe absolument vertigineuse, je le dis, l'Insee estime entre 20 et 25 milliards d'euros pour une année de fraude à la TVA pour contribuer à sa fiabilisation la DGFIP a initié, environ 500 contrôles aléatoire en TVA dont les premiers résultats sont attendus pour le dans les prochaines semaines, évidemment je transmettrai au Parlement, de plus, la loi de finances pour 2020, a permis d'augmenter l'arsenal juridique disponible et la coopération entre administrations et facilité par l'ouverture ou l'accès croisé aux applications, notamment pour lutter contre la fraude à la TVA à l'importation dans ce PLF par ailleurs, nous avons travaillé avec le Parlement, plusieurs mesures qui nous donne de nouvelles armes, réforme de la procédure de suspension des numéros de TVA intracommunautaire, élargissement des compétences des officiers fiscaux judiciaires à l'escroquerie à la TVA, sur un plan opérationnel, la DGFIP a également engagé des actions spécifiques en ciblant des secteurs à risque par exemple l'utilisation abusive du régime de TVA sur la marge dans le secteur du négoce des véhicules d'occasion ou s'agissant des Roussel la judiciarisation précoce des dossiers détecté par l'administration par l'administration fiscale, je vois, madame la présidente, que j'arrive au bout de dix minutes il me reste une page, je peux la finir où c'est vraiment minuté. C'est ces minutes et c'est assez rare, les moments où nuitées pour le gouvernement, ben alors ce que donc quel pays vous pouvez vous pouvez la résumé, je suis sûr que Vladimir très bien non mais sinon ce que je peux faire, c'est la la terminer en répondant sur le premier amendement

Donc, surtout, les travaux sont engagés pour une transparence accrue des transactions assujettis à la TVA à partir de 2024 grâce à une meilleure maîtrise de la donner, d'une part, cela veut dire que débutera auprès des plateformes électroniques, la collecte des données relatives aux opérations réalisées via leur MarketPlace, d'autre part, grand chantier dont nous allons beaucoup être amené à reparler ensemble ici la facturation électronique se déploiera dans les relations entre assujettis à la TVA à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, ça arrive très vite, l'ensemble de ces mesures doit contribuer à sécuriser les ressources de l'ensemble des bénéficiaires de la TVA à un horizon proche, oh la la seule TVA je vous rappelle que la performance du contrôle fiscal continue de s'améliorer, le montant des droits rappelés en 2021 est égal à 13,4 milliards d'euros, c'est 5,2 milliards de plus que 2020, 2020 était une année particulière, c'est 1 virgule 7 milliards de plus qu'en 2019 le contrôle fiscal se transforme, nous faisons plus de prévention, nous ciblons mieux les contrôles en fonction des risques, notamment grâce aux Data Mining en 2021, la part des contrôles issu du Data Mining 45 % contre cible à 40 enfin concernant les remboursements à des politiques publiques et j'en termine là, madame la présidente, je souhaite rappeler que la suppression de la contribution à l'audiovisuel public est une mesure nationale qui permet de supprimer un impôt injuste car forfaitaire due par de nombreux ménages modestes et aisément contournable et obsolète, en maintenant la même ambition du financement du service public de l'audiovisuel, s'agissant du crédit impôt recherche, je veux rappeler que ce dispositif a pour objectif de stimuler les investissements des acteurs privés en recherche et développement, il s'agit d'une dépense fiscale très importante pour le budget de l'État mais aussi un des dispositifs les plus au coeur de l'attractivité économique de notre pays, je termine très rapidement, c'est la toute fin, sur la suppression de la CVAE, l'enjeu est de poursuivre la baisse de la fiscalité de production en supprimant intégralement l'impôt qui génère le plus d'effets économiques néfaste à la compétitivité des entreprises françaises, j'ai bien conscience que cette assemblée a rejeté l'article 5 en première partie, ça ne m'a pas échappé comme j'ai eu l'occasion de le dire le gouvernement regrette fortement cette décision, je ne convaincrai sans doute pas une majorité d'entre vous, mais je veux néanmoins redire que nous en avons besoin pour la souveraineté industrielle mais on nous aurons l'occasion d'en reparler dans les amendements puisqu'un amendement et la traduction concrète de l'absence de suppression de la CVAE merci et désolé encore pour les deux minutes. Bien, nous allons maintenant procéder à l'examen des amendements sur la mission Engagements financiers de l'État ne commençons par le onze 443 monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Si madame la présidente, en fait de ici on s'est largement exprimé sur le le c'est-à-dire le cantonnement dans un programme de la dette Covid donc on va dé-cantonné on était contre le cantonnement, donc on va pouvoir vous proposez de supprimer le programme et donc les crédits qui vont avec, en effet, ça mélange un peu les choux et les carottes parce qu'on fait et du capital et des crédits de de de charges d'intérêt, donc ça c'est d'une originalité, Monsieur le Ministre, l'a souligné, donc nous on n'est pas du tout pour une une soupe comme ça je trouve carottes au moment où le budget prend le bouillon, alors je veux bien que ce soir, monsieur le Ministre de la pédagogie, mais ce n'est pas le budget de l'Éducation, Merci beaucoup, c'est un avis défavorable, la crise a pesé sur notre endettement, l'objectif de dispositifs, c'est de pouvoir identifier retracer suivre l'amortissement de la dette liée à la crise pendant la crise Covid nous avons parer au plus urgent, mais maintenant que nous sortons de cette crise sanitaire, nous devons rembourser cette dette, c'est par la croissance que nous rembourserons cette dette notamment chaque année une partie du surcroît de recettes liées à la croissance est affectée au remboursement de la dette Covid de l'État avec ce programme, il s'agit de pouvoir dire chaque année d'ici 2042 la hausse de la dette estimée fin 2021 était de 165 milliards, voilà où nous en sommes du remboursement de la dette de l'État, lié à la crise Covid je crois que c'est un enjeu de lisibilité et de transparence sur la gestion de nos finances publiques de responsabilité aussi et je crois que ça correspond à une attente des Français qui, évidemment, et beaucoup de questions sur cette dette Covid et ça permet d'avoir les choses de manière lisible et transparente. Et cet amendement propose de remettre un peu, je veux dire la sincérisation la cohérence dans les prévisions du gouvernement, soit on croit aux hypothèses et de toute façon, c'est très difficile aujourd'hui de faire des hypothèses économiques et macro économique, celui qui a de bons résultats, c'est il gagne au Loto, ce qui est certain, c'est que nous avons est supprimé 2 milliards de crédits en loi de finances rectificative ce matin pour les les PGE et là je suis propose étant donné lois d'écoulement et la suppression sur le le les garanties d'État de diminuer de 700000

soit l'hypothèse de pour les entreprises et ben, elle va être bien bien pires, parce qu'elles vont toutes prendre le bouillon, comme je l'ai dit tout à l'heure parce que il y a des crises de l'énergie, et c'est ce qui nous disent : si on prend le bouillon, c'est pas les PGE c'est les Urssaf d'abord et la crise de l'énergie, donc nous on essaie d'être cohérent, soit vous croyez vos dispositif de garantie des entreprises, et cetera et à ce moment-là, tout ira bien et à ce moment-là, c'est des prévisions et trop tout, donc nous l'avons mise réduites de 700 millions d'euros. L'avis du gouvernement. C'est évidemment un avis défavorable, on a besoin de ces crédits. Pour pouvoir rembourser les entreprises on a tenu compte de la sinistralité des entreprises et on ne peut pas comparer ce qu'on prévoit pour 2023 avec le montant des crédits qu'on a annulé en 2022, quand on voit les aléas bien plus grave pour 2023 que ce que nous avons connu en 2022, donc c'est un avis défavorable je ne voudrais pas y voir un moyen simple pour la majorité sénatoriale de faire des économies dans le PLF on a beaucoup parlé au moment de la fin de la partie, hein, du fait qu'à l'issue de l'examen de la partie, hein, il y a un seul de 4 que dans la loi de programmation des finances publiques, vous vous êtes engagé un solde de quatre six ce qui nécessite un montant de 10 milliards d'euros d'économies, j'ai vu qu'hier vous aviez annulé un milliard sur la dotation pour imprévisibilité et accidents, c'est un milliard facilement trouver de ce point de vue-là du tableau à la fin, là il y a 700 millions. Reste à peu près 8 milliards à trouver mais je pense qu'il faut les chercher plutôt dans du structurel voilà. Merci Madame Goulet, Goulet, le président, je suis, je suis désolé pour le rapporteur, mais celui-là, je ne peux pas le voter parce que le risque que court toujours donc vous, vous ne pouvez pas supprimer des des fonds alors que le risque existe toujours c'est c'est le c'est le principe de de cette ligne budgétaire, donc cet amendement là moi je peux pas le voter. Sur cet amendement, il y a une demande de scrutin public du groupe, les républicains, je rappelle que cet amendement de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin clos vous pouvez laisser les cartes dans les terminaux parce qu'il y a un scrutin public ensuite sur le la mission. Votants : 343 exprimés 225 pour deux cents contre 225 l'amendement et donc adopté, nous passons maintenant au vote des crédits de la mission. De nouveau scrutin public, toujours à la demande du groupe, les républicains, le scrutin est ouvert.

crédits sont adoptés, nous passons maintenant à l'examen des crédits participation financière de l'État figurant à l'article D l'amendement 441 au nom de la commission des finances, monsieur le rapporteur. Oui, c'était avant Monsieur Husson et dans la commission des finances, il tire la conséquence pour le CAS PFE participation financière de l'État de du vote que nous avons exprimée juste avant, en supprimant la dette quand Covid cantonné, c'est juste la traduction et la cohérence, un amendement de cohérence. Monsieur le ministre. Avis Avis cohérent ben en cohérence avec mon premier avis défavorable sur cet amendement qui, qui est liée immédiatement au premier. Donc, au moment de la Commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, je mets au vote les le compte spécial participations financières de l'État qui est pour, qui est contre. Elle est adoptée, j'appelle maintenant les amendements rattaché au crédit du compte spécial participations financières de l'État, on commence avec un amendement 105 de monsieur Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, cet amendement, demande au gouvernement d'élaborer un rapport d'évaluation je sais l'attachement comporte 6 rapports sur la disposition adoptée dans la loi de finances rectificative pour 2020, qui conditionne la prise de participation de l'État, via l'Agence des participations de l'État dans une grande entreprise à la souscription par cette dernière d'engagements en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en l'état la disposition adoptée ne concerne que les prises de participation via l'APE débloqués dans le cadre du plan de relance, soit seulement 2 entreprises un tel rapport vise à étudier l'opportunité des conditions d'un élargissement et d'une pérennisation de la mesure pour les les prises de participation de l'État, via l'APE au-delà du plan de relance et son élargissement à d'autres types d'aides publiques, en particulier aux prises de participation via Bpifrance par ailleurs, ce rapport devra évoluer évaluer la pertinence des engagements demandés aux entreprises et leur éventuel renforcement notamment un élargissement du périmètre des missions concernées de sorte à couvrir les activités des entreprises à l'international, ainsi que la mise en place éventuelle de sanctions en cas de non-respect des objectifs fixés. identique madame de la Drees compta merci madame la présidente, très bien défendu par mon collègue, je vous remercie, quel est l'avis de la commission. L'avis de la commission et d'une demande de retrait, d'abord parce que le dispositif qui est proposée par les amendements fait référence au crédit du plan de relance qui aurait abonder le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'État, or aucun crédit de la mission, plan de relance n'a été voté en faveur du casse, qui a eu recours uniquement aux crédits voté dans l'urgence de la première vague de l'épidémie de Covid 19, soit bien avant elle, la politique de relance décidées par le gouvernement, ensuite, ce qui ne semble pas utile de demander un rapport au gouvernement sur des éléments qui sont de toute façon, rendu public par les entreprises elles-mêmes, en effet, l'article 66 de elle fr prévoit la publication d'un rapport annuel des entreprises sur leurs engagements climatiques. Monsieur le ministre. C'est une proposition de retrait parce que, en fait, le rapport que vous demandez au niveau de l'État, il a été publié il est disponible sur le site de l'APE sur la mise en oeuvre de l'écho d'ici à une éco-conditionnalité en général après, vous avez des rapports qui sont publiés chaque année par les entreprises sur le respect de leurs obligations et ça vous le trouvez dans les dans les déclarations extra-financière des entreprises, donc en fait c'est satisfait. Il est retiré, madame, aussi il est retiré, nous passons donc au au vote des crédits du compte spécial Accords monétaires internationaux qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté ensuite le vote des crédits du compte spécial Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics, la commission a émis un avis favorable à la de et crédit qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés, nous procédons l'examen de l'amendement portant sur les crédits de la mission remboursements et dégrèvements figurant à l'article bé, Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour votre amendement 747. Merci madame la présidente, cet amendement procède notamment à l'ouverture de 2,3 milliards d'euros de crédits sur le programme de ce mouvement tire les conséquences de la suppression de l'article 5 que je regrette encore une fois, visant à supprimer la CVAE en ouvrant 2 3 milliards d'euros destinés à la prise en charge par l'État du dégrèvement de CVAE en faveur des entreprises en gros si je résume les choses aujourd'hui, il y a une CVAE qui est payé par les entreprises, mais il y a depuis des années un dégrèvement, c'est-à-dire que pour une partie des entreprises, c'est l'état qui paye la CVAE à leur place et donc, comme il n'y a pas de suppression de la CVAE dans votre copie du PLF on doit remettre les crédits qui des grèves, c'est-à-dire qui permet à l'État de payer à à la place des entreprises, je précise, un point, madame la présidente, en préparant le dépôt de cet amendement aujourd'hui nos services, mais aussi les équipes de la commission des finances du Sénat se sont rendus compte qu'il comportait une erreur puisqu'il que une annulation de crédits 3 milliards, or c'est bien une ouverture de crédit qui est nécessaire pour que l'État prenne en charge ce dégrèvement, à la faveur des entreprises, nos équipes ont ensuite compris que cette erreur qui est évidemment corriger dans l'amendement que je vous présente s'était aussi glissée dans l'article d'équilibre de fin de partie, cela sera rétablie en tenant compte de l'amendement que je vous propose, lorsque vous voterez l'équilibre de parties de ce voilà ce que je voulais signaler et prévenir pour la transparence de vos débats sur la partie de évidemment, alors on a adopté juste hier on se souvient des conditions dans lesquelles l'article d'équilibre, a dû être refait, suite à de nombreuses nouvelles délibérations qui ont été décidées par la majorité sénatoriale pour revenir sur un certain nombre de votes ça entraîné un certain nombre de mouvements de crédit et une erreur s'est glissée

On avait un peu la même question sur ce qu'il y avait des conséquences sur le solde de l'article liminaire : non, vous ne répondez pas, il y a pas, il y a pas de il y a pas d'impact sur OK. Non, il y a un an, pas que sur le solde budgétaire et pas d'impact en comptabilité nationale, c'est bien ça. parfait. Très bien, donc, alors, évidemment, la commission ne s'est pas réuni on le, on le comprend bien, donc on va dire sagesse. Très bien, je mets aux voix cet amendement du gouvernement qui a reçu un avis de sagesse du président de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il être adopté jamais maintenant on voit le les crédits de la mission remboursements et dégrèvements avec avis favorable de la commission sur l'adoption de ces crédits qui est pour, qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés, mes chers collègues, je vais lever la séance, et la prochaine séance aura lieu lundi 28 novembre à 10 heures pour l'examen de la mission Travail emploi du projet de finances, la séance est levée.